La séance est ouverte. Je le garde des sceaux, mes chers collègues. Pour finir le texte ce matin. Bon. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué il y a pas d'observation, le procès verbal est adopté. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023 27 dans la discussion des articles. Nous sommes parvenus à l'amendement numéro 10 au sein de l'article 6, cet amendement en discussion commune le 10 monsieur K navette n'est pas là. Le 60. Toc toc toc. Le groupe socialiste. Le 60 et les membres du groupe socialiste donc. Madame de La Gontrie. Merci monsieur le président. Nous avons commencé à avoir ce débat hier. Concernant la question des des agriculteurs. Nous avons tous été sollicité Je suis élu de Paris, donc vous pouvez sourire. Mais il y a des agriculteurs à Paris. Mais néanmoins. En tant que porte-, parole de mon groupe, tous mes collègues ont été sollicités et les agriculteurs ont manifesté une grande inquiétude face à l'élaboration de ce tribunal des affaires économiques parce qu'il. Considère et cela semble exact que l'organisation actuelle est totalement satisfaisante. Donc je pense qu'il faut d'une manière d'une autre, qu'on trouve une une solution et par ailleurs il y a un problème concernant la contribution financière prévue pour avoir accès au tribunal ou à faire des affaires économiques. Je crois qu'il a d'autres amendements sur le même thème. C'est assez choquant de considérer que on exigerait une contribution pour pouvoir à avoir accès au juge. Sachant qu'il existe dans notre droit des. Possibilités de condamnation pour procédure abusive et cetera et cetera donc. L'accès à la justice ne peut pas être, il est déjà coûteux mais ne peut pas être officiellement payant. Donc c'est pour cela que nous avons déposé cet excellent amendement de mon collègue Sébastien Pla qui est. Malheureusement, retenu par d'autres obligations comme on dit. Merci. Le 270 du gouvernement, monsieur Merci monsieur le président. Cet amendement a pour objet de maintenir les procédures amiables et collective des professions réglementées du droit au tribunal judiciaire. Ce transfert du contentieux des procédures collectives des professions réglementées du droit au à eux a été envisagée un temps par le groupe de travail sur la justice économique avant d'être écarté et, au terme de nos consultations. De l'été dernier et de cet Automne. Nous avons également écarté cette solution pour, pour 2 raisons. D'abord les professions du droit hein n'exerce pas au sens strict, une profession à caractère économique. Et l'autre raison de cette exclusion c'est de garder au sein du tribunal judiciaire. L'ensemble du contentieux qui concerne ces professions du droit. Merci. Monsieur Bena Roche vous nous présenter les 200 et 164. Tout à fait monsieur le président. Alors ce qui concerne de choses que que j'avais présenté en commission qui est, qui est celui que présente ici Joël Labbé. Cet amendement fait je touche le monde agricole comme comme on l'a dit tout à l'heure, je rappelle que aujourd'hui des procédures collectives agricoles sont au nombre de 1200 par an et que sur ces 1200 il y a 46 pour % traités par les tribunaux judiciaires 46% aboutissent à des liquidations judiciaires alors que le taux aujourd'hui au tribunal de commerce toutes procédures confondues est de 70%. Ça c'était pour rappeler le contexte et. Le monde agricole, on le sait à de fortes spécificités qui nous font penser que cette expérimentation en dehors de ce que je viens de dire est inadapté. Le système en place aujourd'hui avec la compétence du tribunal judiciaire. fonctionne plutôt bien, même s'il peut être amélioré. D'après les retours que nous avons des différents. Syndicats agricoles, les délais sont convenables. La procédure permet l'accompagnement des agriculteurs pour maintenir les exploitations et le taux de liquidation judiciaire reste du coût relativement faible. Par ailleurs la filière agricole est très petite. Ce qui entraîne une très forte. Inter connaissance on va dire entre dans ce monde, ce qui pose problème pour la neutralité de la justice avec le système proposé. Il y a aussi la spécificité du foncier qui entraîne en local, on le sait, beaucoup d'enjeux et parfois des conflits qui peuvent poser des questions quant au fait qu'un agriculteur soit jugé par ses pairs et pas par le tribunal judiciaire. Par ailleurs, le ciel les risques psycho-sociaux sont très fort d'agriculture plus que dans les autres professions. On a vu le taux de suicide chez les agriculteurs et qu'il est très difficile pour un agriculteur, de ce fait de parler à leur père lorsqu'ils sont en difficulté la formation au tribunal judiciaire reste dans l'enceinte du d'assistance extérieure au monde agricole les agriculteurs donc ouais d'appréhension. Alors que cette profession connaît un très fort taux de mal-être au travail de suicide déstabiliser les procédures collectives à Paris bien peu au portent l'APCA exprimé dans une audition au Sénat en 2021 sur d'opposition à ce transfert. Âge. Je croyais que vous aviez fait une défense commune des deux puisque c'était un amendement de repli le deuxième mais allez-y. Ah oui. Non mais c'est pour ça que je lui laisser un peu plus de temps mais bon. Monsieur Bénard au chalet.

On y va alors cet amendement de repli propose un échevinat systématique pour le secteur agricole. La taille de la filière L la agricoles étant très réduite. L'échevinat je permettrait de garantir une neutralité. On l'a vu et une indépendance des Césaire au bon fonctionnement de cette juridiction. Le secteur agricole. Qui est caractérisé par les risques de conflit que je viens d'évoquer. Fait qu'il est en effet probable que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés aux futurs ce qui expliquerait et ce qui impliquerait des risques d'absence de neutralité lors des jugements pour d'autres agriculteurs. Nous proposons donc que la formation de jugement pour le secteur agricole soit présidée par un magistrat du siège. C'est un Volvo propose pour compléter les garanties sur l'absence de conflits d'intérêts que soit respecté le principe du pluralisme syndical dans la désignation des assesseurs. Les formations de jugement. Assis. 2 assesseurs issus de 2 syndicats agricoles représentatifs différents cela limiterait le risque de conflit d'intérêts via une représentativité élargie du monde agricole au sein des formations de jugement. Merci cher collègue donc je confirme que le 169 et de 82 ne sont pas défendus et je veux l'avis de la commission sur les quatre amendements le 10. Merci monsieur le président. Pardon le 60. Sur le 60. Oui, donc sur le 60. Madame Le de La Gontrie. De choses. le fait que. Il y a une contribution, c'est l'article 7. Donc, nous en parlerons tout à l'heure par contre. Non aux agriculteurs. Comme je l'ai dit hier, la Commission a essayé de répondre aux inquiétudes des agriculteurs en incluant des agriculteurs des d'expérimentations au sein des juges consulaires ensuite par rapport aux craintes possible. Déjà, je voudrais dire que sur les baux ruraux les agriculteurs siège déjà. Et visiblement ça se passe pas si mal que ça donc un agriculteur, par définition, n'est pas forcément malhonnête et par ailleurs, non mais c'est un peu la petite musique qu'on entend, il y a des problèmes de territoire et puis on a des inquiétudes. Donc moi je pense que non. Ça n'est pas on n'a pas à se penser comme ça et. Que par ailleurs il y a des règles de déport très clair, c'est une expérimentation, regardons comment ça fonctionne. Mais a priori, quand vous dites les agriculteurs, ça n'est pas tout à fait juste une association effectivement nous a construit contacté solidarité paysanne. Madame de La Gontrie. Vous plaisantez parce que vous étiez de Paris solidarité paysanne et du 93, on peut tout aussi s'interroger sur la vraie ruralité. De de cette association. Non, mais qui défend effectivement plutôt des très petits agriculteurs. Je crois qu'. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans les tribunaux de commerce, ils savent accompagner aussi les petites entreprises et l'accompagnement sera probablement plus fort encore, parce que là cette association accompagne des petits agriculteurs mais pas tous les tribunaux de commerce seront s'occuper de tous. Donc il me semble que tous ces toutes

mais ça leur arrive pour autant. Sachez que c'est une position constante du Sénat que d'inclure l'ensemble des professions vous incluez là dans cette expérimentation aussi les associations, l'ensemble des professions libérales, objectivement il n'y a pas de raison que les professions réglementées du droit en soit exclus de la même façon, effectivement on pouvait dire que, attention, ils ne pourront pas siéger nous précisons bien que ils ne siégeront pas évidemment dans le ressort dans lequel ils exercent mais ils peuvent tout à fait siéger à côté. Et donc du coup ils pourront être jugés par leurs pairs pas leur père concurrents mais leur père malgré tout. Le 211, bah c'est de nouveau les agriculteurs je pense y avoir répondu et ensuite. Quant à Monsieur Bénard Roche pour le 164 qui propose que l'on mette un magistrat professionnel. Je crois que nous y avons répondu aussi une grosse inquiétude de tous les tribunaux des des futurs tribunaux des affaires économiques et des actuels, tribunaux de commerce qui refuse toute échevinat je donc je crois que c'est pas la peine de, des, de les provoquer en en rajoutant donc défavorable avant. Oui j'ai j'ai compris vis du gouvernement sur les trois amendements en dehors de celui du gouvernement naturellement. Président mais vous avez tout résumé. Je suis débat fort défavorable à tous les amendements. Naturellement, je suis favorable à l'amendement déposé par le gouvernement. Je veux rappeler que ça ne concerne pas que les avocats mais aussi les notaires, que les notaires sont des officiers publics. Et. J'entends bien, mais nous il nous semble qu'ils doivent être rattaché au tribunal judiciaire. C'est le sens de cet amendement j'entends que la commission ne partage pas, à mon avis et c'est bien son droit. Voilà monsieur le président, ce que je veux redire mais très très brièvement, c'est que. D'abord tous les agriculteurs ne sont pas défavorable à cette réforme. Ça n'est pas exempt de le dire ainsi. Et l'idée, c'est justement de les mieux protégées. Parce qu'il y a peu différence au fond entre une petite exploitation agricole, une petite entreprise. Et nous avons des juges qui sont spécialisées et puis. L'autre idée naturellement c'est que toutes les mesures qui sont prises en amont et qui permettent de sauver des petites entreprises. Et ben justement. Elles doivent s'appliquer et mieux s'appliquer aux agriculteurs. Vous avez rappelé le nombre impressionnant de suicide dans le monde agricole et je pense que mieux les protéger devrait nous convaincre tous d'adopter cette réforme. Merci. Je précise tout de suite. Attendez monsieur Bena. Que je suis saisi d'une demande de scrutin public par la commission des lois sur l'amendement numéro 270 du gouvernement. Et nous aurons l'occasion de le faire. Mais monsieur Bena Roche. Explications. Merci monsieur le président. D'abord je voulais répondre à la rapporteure que si elle a entendu une seule fois dans ma bouche. Des paroles qui mettait en cause l'honnêteté des agriculteurs. Faudra m'les préciser parce que d'aucuns cas ce n'était la réalité de mes propos.

et par ailleurs je n'ai pas entendu madame la rapporteure de soutien franc alors c'est pas tous les agriculteurs, vous avez raison monsieur le ministre de Madame la rapporteure. J'ai pas entendu dans plus beaucoup d'agriculteurs y compris la FNSEA qui a défendu ce projet. Par ailleurs, quand vous dites qu'on va améliorer la situation. Aujourd'hui je n'ai pas non plus entendu beaucoup d'agriculteurs qui ont dit que le système en place était un système qui ne fonctionnait pas. Je comprends très bien qu'on veuille rénover ou modifier un système qui ne donne pas satisfaction à la majorité mais c'était pas le cas. Ensuite monsieur le. Garde des Sceaux quand vous dites que du coup ça va mieux les protéger. Je l'ai rappelé. En préambule, aujourd'hui les taux d'entreprises qui. Finissent en liquidation. Après passage au tribunal de commerce est beaucoup plus important que celui d'agriculteurs après passage au tribunal judiciaire. Donc est-ce que pour autant ça va améliorer là d'un seul coup, je ne vois pas quel réseau améliorer ça et l'élément que je donnais c'était pas un élément de mise en cause de l'honnêteté. C'était un élément qui faisait qu'effectivement y compris au niveau psychologique, il est très difficile. Un agriculteur de passer devant ses pairs. si on est si on le fait passer devant ses pairs, ça complexifie les choses et ça risque au contraire d'amplifier le problème donc je voulais répondent à ces arguments qui me paraissent pas justifiés. Merci monsieur Bonnecarrere. Oui 2 volets, le volet agriculteurs le volet professions réglementées sur deux volets, agriculteur. Je crois que la future compétence, du moins à titre expérimental des tribunaux d'affaires économiques. Pour le monde agricole sera une évolution favorable, et en particulier. Pour les agriculteurs les plus modestes pour 2 raisons, la première c'est que dans les. Le fonctionnement de notre judiciaire sauf peut-être les plus importants l'activité procédure collective est une une activité très à la marge peut représenter une demi-douzaine de dossiers par an, autrement dit la technicité des tribunaux judiciaires en matière de procédure collective est à mon avis a beaucoup relativisée par contre les tribunaux commerces ont une forte expérience, il a en particulier une expérience de la prévention de la négociation. Les tribunaux de commerce sont une obsession si vous ne méritez la formule que les difficultés du monde économique soit connu en amont de la sieste le plus en amont possible de telle manière que les préoccupations du monde agricole et en particulier des plus modestes se rend à mon avis fort bien fort bien pris en compte en ce qui concerne la question des professions réglementées. On peut dire effectivement les 2 choses, il y a une tradition pour les professions réglementées, d'être dans le monde. De des tribunaux judiciaires de la chancellerie de la chancellerie, on peut observer. Que si l'objectif est d'ouvrir le monde de la justice également le monde judiciaire il me paraît. Assez cohérent de les intégrer avec les autres professionnels. Le vrai sujet en particulier sera celui des notaires, ils ont une obsession, ne pas être pris dans le droit commun. Vous savez que le mot autorité de la concurrence, depuis la loi Macron et tu. Un mot qui crée un particulière agacement dans la profession notariale et que ils ont une crainte à travers une banalisation à travers les tribunaux affaires économiques de-ci mais nous avions pris position en sens contraire. Je vais mettre aux voix, donc je vous rappelle que sur le 270 sur un scrutin public. Le 60 d'abord avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté le 270 donc scrutin public. À la demande de la commission des lois, avis de la commission défavorable à du gouvernement par définition favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56, le scrutin est ouvert.

Sur l'amendement votants 343 exprimés, 252 pour 39 contre 213. L'amendement n'est pas adopté. Le 211 avec 2 avis défavorables qui. Pour. Qui est contre. Rejetée même vote pour le 164. Même vote rejeté. Je passe au 271 du gouvernement, monsieur le garde Merci monsieur le président. Je voulais qu'on maintienne le traitement du contentieux des baux commerciaux au sein du tribunal judiciaire. Sauf lien de connexité avec. La procédure collective. Je rappelle simplement que l'extension de la compétence du TA eux. À tous les baux commerciaux ou autres convention n'est pas conforme aux conclusions des états généraux de la justice. Je vous enfin dire que nous avons vu évidemment des échanges avec des représentants. Du monde agricole à la fois. Lors du groupe de travail et de l'élaboration des des mesures que nous avons reprises mais également à mon niveau lors de l'élaboration du projet. Ces consultations sont d'ailleurs pas terminée parce que au moment de préparer les décrets nous rencontrerons évidemment tout le monde. Merci avait de la commission. Défavorable. Je ne sais pas. Oui, monsieur le président. Je ne sais pas si c'est contraire au. Au à la vie des états généraux de la justice mais par contre c'est totalement conforme aux propositions faites par le Sénat au cours des dernières années. Cette réforme de notre point de vue a le mérite d'assurer une meilleure lisibilité pour les justiciables. Ce qui relève du commerce à. Et et du monde économique vont au tribunal des affaires économiques. et donc ça permet une meilleure. Cohérence et répartition des compétences entre tribunal judiciaire et tribunal des affaires économiques, on arrête de se poser la question si on relève du tribunal des affaires économiques. Alors y compris pour nos beaux nous allons au tribunal des affaires économiques. Au surplus les baux commerciaux sont par essence un domaine exclusif de la vie des affaires, qui a paraît donc naturel de confier à la juridiction spécialisée en la matière. Merci. Mais on voit le 271 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est. Pour.

Le l'intégration du secteur agricole dans les tribunaux des affaires et. Que nous venons de voter, alors le premier le 162 a pour objectif d'assurer une protection maximale du secteur agricole matelas qu'il est. Intégré dans l'expérimentation des tribunaux des affaires économiques. Malgré que le système actuel soit suffisamment rapide et permettez un accompagnement des agriculteurs et. À via ce problème de l'Iliade atterré qui a rien à voir avec une honnêteté ou malhonnêteté supposée. Dans cette profession comme dans les autres d'ailleurs Madame la rapporteure. Les Liens d'intérêt c'est des relations qu'il peut y avoir avec des structures ou des individus qui ont des intérêts dans les décisions qui sont prises, tout simplement. Le conflit a lieu quand l'expert ou le juge risque de prendre une décision qui serait différente si il n'y avait pas ce lien. On considère qu'il y a conflit d'intérêt, dès que les les altère le jugement de l'expert ou sur perçues comme susceptibles de l'être. C'est toute la question de l'intégrité de l'expertise qui est en jeu, l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, relative à transparence de la vie publique définie pour la première fois la notion de conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et les aides et des intérêts publics ou privés qui est de nature à l'affluence est ou paraître influencer l'exercice indépendant impartial et objectif, a une fonction, il convient donc pour nous, que le rapport d'évaluation de l'expérimentation, qui devra être établie. Qui qui est prévu par cet article soient particulièrement attentifs à ces problématiques. D'où la modification que nous proposons. En ce qui concerne le deuxième. C'est un amendement de repli donc le 165, alors attendez. Le 163 c'était oui je veux des défendent le 162 donc c'est celui qui avait pour objectif d'assurer. pomme une prise en compte de la formation des juges consulaires spécifique au monde agricole. Voilà donc ces spécificités et l'importance du secteur et de l'emploi agricole pour les territoires et pour la souveraineté alimentaire. Nécessite une adaptation de la formation des juges consulaires des tribunaux des affaires économiques expérimentaux et enfin le dernier qui est de 165. C'est un amendement de repli qui propose une évaluation spécifique de l'expérimentation pour le monde agricole qui associent les acteurs de terrain via un groupe de suivi permettant d'établir une efficacité supérieure du nouveau tribunal des affaires économiques proposées par le texte. Le système actuel. Qui était celui où les. les. Tribunaux judiciaires se prononcer. Établissait un certain nombre de décisions qui permettait de diminuer le nombre de liquidation. Je l'ai vu tout à l'heure bon c'était rapide et aujourd'hui dans un contexte de mal-être agricole nous pensons effectivement que l'expérimentation qui est menée, doit faire l'objet d'une évaluation spécifique sur. Ce domaine agricole et. Que les travaux d'un groupe de suivi s'associent. Comprenant des acteurs agricoles s'associe à à l'évaluation et permet d'établir entre autres que le taux de liquidation judiciaire et le Mathias de l'emploi agricole a été satisfaisant par rapport au système actuel et que l'impact des nouvelles procédures sur les risques sur les risques psychosociaux en agriculture a été positif. Merci. Avis de la commission sur ces trois amendements. Je vous ai déjà dit qu'il y avait effectivement de toute façon un un des ports. Et des règles de, des ports qui sont obligatoires. Et évidemment ça fera forcément partie de l'évaluation. je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'ajouter des critères. En plus puisque de fait. Je pense que les gens qui feront l'évaluation de regarderont de près. Comment ça a pu se passer et si des conflits d'intérêts trop nombreux et des déports trop nombreux surtout ont ont eu lieu. Concernant la prise en compte du niveau de formation des juges consulaires. Alors pour le coup vous souhaitez les former à la matière agricole mais comme nous avons fait rentrer les juges consulaires, agriculteur. Je pense que cette formation spécifique n'est plus nécessaire et ils iront par contre les juges, agriculteurs se former droit comme tous les juges consulaires et c'est bien normal. Donc il me semble que finalement votre amendement est en quelque sorte et satisfait et enfin quant à la création du groupe de suivi. Alors on comprend bien nous savons que nous sommes des grands brûlés de l'évaluation ici. Surtout à la commission des lois, puisque on a vu des évaluations ne pas arriver au bout et des choses se mettre en place malgré tout. Mais je pense que ça pu servir de leçon puisqu'on le rappelle assez régulièrement au gouvernement pour que cette fois il nous fasse une véritable évaluation avant que l'on mette en place. Et qu'on généralise ou pas. Cette expérimentation. Merci avait du gouvernement sur les trois amendements. Ont été présentés au gouvernement mais je pense que j'ai pas assez des. 10 doigts de mais demain pour les compter. J'y suis défavorable en revanche une évaluation oui au sens d'ailleurs. Qui est donné par le Conseil d'État de ce mot évaluation il est évidemment indispensable que l'on puisse suivre ce que vous avez voté sur la formation des juges et sur les risques. Et les spécificités du secteur agricole, je suis favorable à votre amendement. C'est aussi de nature à rassurer le monde, le monde agricole, il y a un certain nombre de spécificités. Oui. Je pense qu'on peut mieux les prendre en considération et j'entends toutefois le bémol que présente Madame la rapporteure Des. Juges. Consulaires issus du monde agricole. Participeront. Aux décisions, ce qui est être ce qui permet aussi au au monde agricole d'être rassurés. Alors ensuite sur le groupe de suivi. Moi franchement je préfère un échange avec tous les acteurs, dont les parlementaires que vous êtes naturellement. Ça me semble plus fluide, plus simple, plus directe et plus efficace. Donc je suis pour me résumer favorable aux 163 et défavorable aux deux autres, monsieur le président. Hé bien. Je vais les mettre aux voix successivement donc le 162 avec 2 avis défavorable qui. Pour. Qui est contre. Rejeté le 163 avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour.

Merci monsieur le président. L'article 7 qui porte sur l'expérimentation des tribunaux des activités économiques prévoit de mettre à la charge de l'entreprise requérantes une contribution fixée selon un barème défini par décret en Conseil d'État. Cette disposition déroge au principe de gratuité de la justice. En outre, accepter son principe, c'est prendre le risque qu'elle puisse demain être élargie dans son montant et son Champ d'application à d'autres types de litiges. Selon le gouvernement, cette contribution permettrait entre autres de limiter le nombre de recours. Or une telle disposition apparaît inutile dès lors que l'on a déjà constaté une réduction de moitié de l'activité enregistrée par la juridiction commerciale en 15 ans. Il apparaît tout aussi injuste de faire peser sur l'entrepreneuriat privé le financement de la justice alors que le service rendu par les tribunaux de commerce ne sera aucunement améliorée. On rappellera en effet que les juges consulaires sont bénévoles et les Budgets de fonctionnement des tribunaux de commerce en constante diminution. Alors que les charges administratives et les impôts qui pèsent sur les entreprises sont plus élevés en France que dans les autres États européens. Il apparaît inconséquent d'instituer une telle contribution. Faire varier la contribution en fonction du montant du litige frappera plus durement les petites entreprises déjà contrainte d'engager un contentieux lourd. De leur côté, les plus grosses entreprises seront incités à utiliser les règles de droit international privé pour contourner les tribunaux français. Il en résultera une rupture d'égalité devant la justice. On soulignera également l'extrême complexité des critères retenus pour déterminer le montant de cette contribution qui exige le combiné des critères objectifs avec des critères subjectifs. Dans ces conditions le présent amendement propose de supprimer cette disposition qui instaure une nouvelle taxe qui ne dit pas son nom et limite ainsi l'accès à la justice des entreprises vous remercier. Merci Monsieur le Président effectivement tout à l'heure j'avais commencé de de. De traiter ce sujet en fait. On ne comprend pas très bien la logique plus exactement, on voit bien que c'est une logique exclusivement de de recettes. Et donc. J'attire l'attention de nos collègues sur ce que cela veut dire. Sur le reste des contentieux judiciaires, parce qu'au fond pourquoi limiter au contentieux devant le tribunal des affaires économiques, l'idée de la taxation en fonction de, de l'enjeu du du litige Le garde des Sceaux à l'époque avait eu également la même démarche. Je me souviens du combat qui avait été celui d'une partie de de du monde judiciaire contre le principe du timbre qui était imposé pour pouvoir accès aux procédures civiles et qui avait été finalement supprimé. Donc je pense que tout ça et tout à l'heure notre collègue parlait de justice gratuite. La justice n'est n'est pas gratuite. Elle ne l'est jamais. Mais l'accès au juge doit l'être le plus possible, il ne je n'ai jamais il faut en général. Ou souvent avoir recours à un avocat. Vous savez que les conditions d'accès à l'aide juridictionnel sont incroyablement. Restrictive. Et cetera et cetera mais là on affiche la couleur donc je pense que c'est un c'est que nous devons combattre et je dois le dire, Monsieur le Ministre que dans vos vos explications. Rien n'est très convaincant et je le disais tout à l'heure la responsabilisation des partis il y a d'autres moyens

Oui, rapidement puisque le même amendement a été défendu déjà par monsieur Bovary à madame de La Gontrie de poids supplémentaire. Comme c'est dans le cas d'une expérimentation. En fait, de ce fait là, on va avoir une rupture d'égalité entre les justifiable très Net puisque. Dans le dans le courant de la phase d'expérimentation. Selon le territoire national. Le tribunal concerné ou pas.

Le Syndicat des avocats de France m'a fait une remarque qui m'a interpellé quand même. Les personnes morales n'ayant pas massivement droit à l'aide juridictionnelle. Il apparaît que cette mesure sera aussi pour les personnes morales un obstacle accès au juge pour les très petites, les petites et même les les moyennes entreprises ces 2 éléments supplémentaires par rapport à ce qui a été dit, c'est pour ces raisons que nous demandons la suppression de cet article. Merci le 194 monsieur Ouzoulias. Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, je vais pas je

Pardon. Les petites entreprises et louer grosse comme vous voulez. Donc ce qu'on ce qu'on défend, c'est le principe de la gratuité de la saisine de la justice. Je pense que c'est fondamental et là-dessus, il ne faut pas céder. Merci, monsieur le Président R avait la commission sur ces quatre amendements de suppression. Merci monsieur le président. Alors. La Commission pense que l'expérimentation d'une contribution financière pour saisir le tribunal des affaires économiques mérite d'être expérimentée. En 1er lieu, je rappelle que l'accès à la justice n'est pas gratuit. Puisque ne serait-ce que pour faire appel, en matière civile, un timbre fiscal de 225 euros est nécessaire. Par ailleurs il me semble que Madame Taubira elles-mêmes avait mis un timbre au niveau de la justice économique en son temps. Et puis il existe aussi des frais d'avocat si son assistant ses obligations est obligatoire sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mais on sait que nous sommes nombreux à ne pas pouvoir. En 2ème lieu notre commission s'était prononcé de manière favorable au retour d'une taxe introductif d'instance dans le cadre de la mission d'information. 5 ans pour sauver la justice présidée par notre questeur Philippe Bas. la création, la création d'une contribution économique est également une mesure portée par le comité des états généraux de la justice. Enfin cette contribution fera l'objet d'un encadrement strict. Via un barème permettant de s'adapter à la situation économique de la partie demanderesse, le coeur de cible du dispositif étant les litiges d'un montant important de plus de 200.000 euros, ce qui ne correspond qu'à 16% des litiges et des entreprises financièrement solide. Je pense que le gouvernement nous en dira plus. En tout cas lors de son audition. C'est ce qu'il nous a. Indiqué nous avons également proposé un amendement permettant de préciser les critères économiques à prendre en compte en étalant le nombre d'années pour mesurer le chiffre d'affaires en y ajoutant le bénéfice parce qu'on comprend qu'on peut avoir un gros chiffre d'affaires et un tout petit bénéfice et donc il est effectivement important de faire que la prise en compte de cette contribution enfin de de des conditions de la de l'entreprise soit faite pour pouvoir. Être exonérés éventuellement de cette contribution ensuite monsieur barbarie parlait du fléchage effectivement la justice économique. Mais nous le disons et les tribunaux des affaires économiques futures. Auront besoin d'être plus accompagné puisqu'on sait, comme je l'ai dit d'ailleurs. Lors de la discussion générale que la plupart des juges consulaires sont plutôt des mécènes de la justice. Ce fléchage ne peut pas se faire aujourd'hui ce fléchage ne peut pas se faire aujourd'hui dans ce texte de loi, il pourra se faire sur le projet de loi de finances et donc. Nous veillerons au moment du projet de loi de finances qu'effectivement cette contribution soit fléchée vers la justice en général et vers la justice économique en particulier. Donc il me semble que au niveau du sénat alors que nous avons toujours proposé de tester cette contribution. Il me semble. Dommage que nous rejette l'expérimentation, il vaut mieux. Des solutions pour être sûr que ça ne touche pas des entreprises dont nous ne voudrions pas qu'elles en soient victimes mais que nous expérimentions malgré tout quelque chose que nous appelons de nos voeux depuis plusieurs années. Avis du gouvernement. Merci monsieur le président. Monsieur le Sénateur ben arrogent sur la question de la rupture d'égalité je. Vous invite à relire l'avis du Conseil d'État. Il s'agit là d'un motif d'intérêt. Général et il n'a pas échappé au Conseil d'État cette question légitime que vous posez. Il y a répondu. L'idée en réalité elle est mesdames et messieurs les sénateurs, très simple. Il s'agit, à mes yeux. De renforcer l'attractivité du droit. De la. Justice française au moment d'ailleurs où on vient d'installer la jupe juridiction unifiée des brevets, l'attractivité de la place de Paris est en cause et pourquoi et les états généraux l'explique parfaitement bien de façon très curieuse paradoxal peut être même incompréhensible. Les acteurs économiques disent que la justice néerlandaise allemandes, anglaises. Est meilleur que le nôtre parce que c'est justice sont payantes, c'est curieux c'est le syndrome de la marque. C'est-à-dire que vous avez un costume et puis un autre, c'est exactement le même tissu la même facture. L'un porte une marque l'autre pas, certains préfèrent la marque, c'est comme ça je n'y peux rien. Le rapport des états généraux sont extrêmement explicites sur ce point. Alors maintenant c'est le sénateur babary je j'en j'entends vos arguments. J'entends vos préoccupations. Sont aussi les miennes, je le dis et je le redis, la contribution économique. Dont je souligne une fois encore le caractère expérimental. Ne sera due que par les grandes entreprises et pour les litiges les plus importants. C'est la raison pour laquelle, avant même que les barèmes ne soit défini par décret. Nous avons mis en place de sécurité. La première, un mode de calcul qui tient compte du montant de la demande de la nature du litige et de la capacité contributive de la partie demanderesse, et ce dans la limite de 5% du montant du litige plafonnés à 100.000 euros 2ème sécurité une exonération systématique pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Les procédures amiables ou collective et les personnes morales de droit public. Je souhaite évidemment être à votre écoute, car à travers vous ce sont les craintes de nos concitoyens petits entrepreneurs, petits patrons qui s'exprime et voilà ce que je propose, afin de répondre à vos préoccupations et de sécuriser davantage notre dispositif. Je propose une 4ème cause d'exonération de contribution pour les entreprises de moins de 250 salariés. Comprenez donc. Votre amendement. Vise à défendre. C'est un clin d'oeil que je vous adresse naturellement les grosses boîtes. Voilà et tout le monde l'aura noté. Bon ce seuil des salariés un ce que nous connaissons bien, il a le mérite de la clarté. Et qui en lien Direct d'un point de vue constitutionnel avec l'objet de la contribution ça. C'est extrêmement important. Voilà ce seuil pour qu'il s'applique pleinement et atteignent notre objectif. Il devra concerner évidemment tous les demandeurs personne physique ou morale. Quelle que soit la nature de leur activité. Merci. Monsieur Bonnecarrere. Explications de vote. que l'on retrouve tous les 10 ans et qui a passionné le monde judiciaire à travers le droit de timbre installé puis supprimée pour les hein. La justice et par principe, gratuite pour les autres. Ah la hein coûte dans une société démocratique, il faut que ceux qui ont les moyens d'accéder à ce service. Hé bien participent à son financement et ceux qui n'en ont pas les moyens, bénéficient de la solidarité nationale à travers l'aide. Juridictionnelle. J'avoue ne plutôt sur la seconde. Opinion d'autant plus que. Il y a quand même l'idée me semble-t-il de d'avoir une prévention de ce qui pourrait être un contentieux de mars mais l'argument peut être le plus décisif. En faveur de la position de la Commission et. Du projet du gouvernement, c'est de savoir si on veut vraiment donner une chance à l'amiable. Si vous voulez vraiment privilégier l'amiable dans ce pays. Il n'y a pas d'autres me semble-t-il d'autres solutions que de dire à notre ont nos concitoyens que la justice a effectivement un coup et que s'il y a une procédure. En tout cas devant le tribunal des affaires. Des Cela se traduit par une participation aux frais et cela repose à mon avis de manière assez pertinente. Une sorte de priorité à la conciliation dans ce type de District. Il faut les raisons pour lesquelles nous serait sont tout à fait aligné la position exprimée par la Commission mais. Monsieur Barry. Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, j'entends bien que s'il s'agit d'une position traditionnelle du Sénat. Encore faut-il, tenir compte de la situation et du calcul de la contribution. Qui elle. N'a pas été pris en compte. Si on fixe cette contribution en fonction de la capacité financière du demandeur. Si c'est une grosse entreprise qui est en différents avec une petite entreprise et que c'est la petite qui perd. Elle devra dans les dépend payer le montant de la contribution qu'aura. Qui aura été calculé pour demandeurs donc. Ce calcul là. Doit remettre en cause la vision traditionnelle du Sénat sur la contribution. En question. Monsieur le monsieur le ministre. À la fois votre remarque est est légitime. Et pertinente mais il faut évidemment veiller qu'il ne s'agisse que de litige entre grandes entreprises, évidemment le but non mais moi je, je dis que cette contribution. Expérimental et très utile pour l'attractivité de la place de Paris en matière économique. J'entends vos réserves et j'entends co-construire avec vous certains nombres de remparts nous permettant d'avoir des certitudes et de ne pas franchir. Effectivement ces écueils que très justement vous. donc construisons ensemble ces écueils. Ses frontières. Il s'agit pas évidemment. Qu'au sortir du tribunal. Des activités économiques, une petite entreprise soit démoli. Ça n'est. Attends rien le but. Mais quand vous avez des contentieux qui durent 5 6, 7 ans, parfois dilatoires qui mobilise la justice qui mobilise tous les acteurs des juges consulaires qui interviennent gracieusement, il faut le dire et leur rendre hommage. Pardon de vous dire qu'il n'est pas injuste et qu'il n'est pas indigne que l'on envisage effectivement une contribution à nous ensuite dans de la co-construction parce que au fond. On peut avoir les mêmes préoccupations et nous avons les mêmes préoccupations à nous ensuite de construire ce qui permet de protéger évidemment les plus faibles qui méritent de l'être. Brièvement avant le vote. Madame la rapporteur. Merci monsieur le président. Oui. Monsieur. Bonnecarrere a a raison et j'aurais dû le souligner, il est vrai que si on va vers l'amiable. on n'est pas assujettis à cette contribution, donc c'est effectivement important pour pouvoir développer l'amiable. Ensuite monsieur Babary, vous avez raison, le dispositif n'est pas parfait et c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend le barème et on souhaite le voir. Cela dit, je voudrais attirer votre attention sur le fait que si nous ne le vote, ont pas là. Nous n'aurons à mon avis, aucune chance de pouvoir modifier le dispositif. Donc ce que je vous propose c'est de voter le principe éventuellement. D'amender derrière. À travers puisque je sais qu'il y a des, des amendements qui qui vont venir de l'amender de le retravailler mais le faire faire. Simplement sauter l'article aujourd'hui c'est ne pas donner du tout de chance. Ah cette contribution de pouvoir être expérimenté. Merci. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur les quatre amendements identiques de suppression. Je vous rappelle que la commission et le gouvernement sont défavorables. Il va être procédé au scrutin public conformément à l'article 56, le scrutin est ouvert.

Votants 342 exprimés, 339 pour les amendements de suppression, 97 contre 242. Ils ne sont pas adoptés et je passe à l'amendement Monsieur air oui je vous en prie. Merci monsieur le président. Donc. Cet amendement là de notre collègue Jean-Yves Roux est assez simple. Il vise à prévoir que seuls les litiges supérieurs à 500.000 euros seront assujettis à la contribution financière prévue à l'article 7 donc du projet de loi. Avant tout, nous tenons à rappeler notre attachement au principe de gratuité de la justice, mais nous entendons que tout principe connaître des dérogations et en particulier pour les procès commerciaux et largement économiques opposant des entreprises. Seulement, nous considérons qu'instituer une telle contribution sans distinction. Montant des litiges risque de pénaliser par exemple certaines petites entreprises aux moyens modestes. Monsieur le Ministre, parlait de rempart. À mettre en place, hé bien nous y contribuons. Merci. Avis de la commission. je pense que l'idée là c'est vraiment de retravailler le dispositif donc défavorable pour l'instant mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire d'ici l'issue de ce texte. Merci avait du gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président, ce sénateur. Moi je ne peux pas dire que je sois défavorable. On veut mettre un certain nombre de de de de seuil. Je dis que c'est un peu prématuré, puisque dans la cohérence avec ce qui a été dit précédemment, je vous propose un, un retrait on on travaille sur ces questions, on essaie de.

Merci monsieur le président. Chers collègues, en fait nous avons déjà réintroduit en commission la notion de bénéfice. Pour justement amenuiser simplement le chiffre d'affaire puisqu'on sait qu'on peut avoir un gros chiffre d'affaires et un tout petit voire un bénéfice nul ou négatif. Malheureusement. Donc je pense que votre amendement est satisfait. Avis du gouvernement. Si Monsieur le Président une supplique. Monsieur le sénateur voulez pas le retirer puisque c'est la même logique est la même cohérence. On y travaille et puis. Ensuite, on affine. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avons appris avec beaucoup d'émotion la terrible attaque par un individu armé d'un couteau contre plusieurs personnes dont des enfants dans une aire de jeux à Annecy. L'individu a pu être interpellé grâce à l'action rapide des forces de l'ordre mais il y a plusieurs blessés parmi les enfants dans des conditions extrêmement grave avec un pronostic vital engagé. Au nom du Sénat tout entier. Je souhaite exprimer tout mon soutien aux victimes et à leurs proches, ainsi qu'aux forces de l'ordre et au secours. Merci. Article 8. L'amendement 233 madame Vogel. Merci monsieur le président. Un peu difficile de prendre la parole après cet hommage. Si vous le souhaitez je vous propose de présenter les quatre amendements à la suite. Je sais qu'ils sont pas dans une discussion commune mais ils sont, ils sont tous liés puisqu'ils sont tous. À propos des des prud'hommes. l'amendement 233, il vise à assouplir les limitations géographiques pour les candidatures pour les prud'hommes. Nous le savons le fonctionnement des conseils des prud'hommes et mise à mal, notamment par un manque désormais chronique de conseillère et de conseillers prud'hommes et les conséquences sont lourdes. D'un côté des délais excessivement longs, il n'est pas rare que 9 mois s'écoulent entre la saisine et l'audience de conciliation qui n'est que la première étape et cela décourage souvent les salariés de saisir les conseils des prud'hommes de l'autre côté on a des prud'hommes surchargé qui croulent sous les dossiers, surtout dans certaines sections. Ceci n'est pas durable et décourage la prochaine génération de déposer sa candidature pour le conseil des prud'hommes. Le problème est donc d'ampleur et certains sénateurs ou sénatrices préconise de renforcer les sanctions contre l'abandon de poste. Nous pensons d'un autre côté, que la solution est ailleurs et que plutôt que de sanctionner nous devrions faciliter les candidatures au conseil des prud'hommes, en particulier des dispositions qui détermine quel salarié peut se porter candidat pour quelle section sont assez strictes car, en règle générale, on ne peut être candidat, que pour le conseil des prud'hommes de son lieu de travail et nous savons que le monde du travail a évolué, notamment depuis le Covid, le télétravail s'est répandu pour certains secteurs, il faut le dire, surtout pour les cadres et 55% des salariés font désormais du télétravail à moins d'une heure par semaine au moins une heure par semaine. D'après l'Insee. Et donc cet amendement. Propose simplement de permettre aux salariés dont le contrat permet de télé travailler au moins 30% de leur temps de travail de candidater au conseil des prud'hommes de leur domicile et non seulement de leur lieu de travail. C'était le 233. Pour le 234. Il s'agit de permettre aux délégués syndicaux d'exercer une fonction de mandataire de listes des candidats de prud'hommes sur leur temps de travail sans texte activités soit décomptée de leurs créditeurs d'syndicaux. Parfois il y a dans le droit des autorisations qui semble a priori accorder plus de liberté, mais qui en réalité se révèle être plutôt une source de contraintes additionnelles dans la pratique et la disposition que nous proposons de supprimer en fait partie. Je m'explique, chaque liste de candidates et de candidats aux élections prud'homales est géré par une ou un mandataire de liste ce sont les mandataires qui doivent collecter les pièces justificatives qui les téléchargent pour déposer la liste qui notifie formellement l'employeur des salariés qui candidate et ce sont encore les mandataires qui reste disponible ensuite pour faire le lien quand parfois des documents manque ou des pièces additionnelles doivent être fournis. Et nous le savons, surtout dans cet hémicycle à un moment où certaines et certains sont occupés à constituer des listes constituées. Cela prend du temps et c'est là où nous venons à un droit qui n'en est pas hein. Actuellement, la loi prévoit que les mandataires de listes qui sont par ailleurs délégués syndicaux puissent utiliser le crédit d'heures dont il dispose au titre de leur mandat pour constituer les listes, nous considérons que c'est un autre travail que de constituer les listes pour les prud'hommes et que ce temps additionnel devait être en plus et non pas imputer au crédit pour ses activités syndicales le 235 maintenant. Le 235 il. Consiste à inscrire dans la loi l'obligation que les formations initiales et continues comprennent des séances sur les procédures de conciliation. Un rapport du Sénat. De nos collègues Canayer de Lattre Gruny. Avait. Fait le constat d'un, d'un manque de formation aux procédures de conciliation, or nous savons que c'est la première étape de de la procédure des prud'hommes et que seulement 8% des affaires sont résolues à l'issue de cette procédure de conciliation. Ce qui est inefficace ce n'est pas l'étape en elles-mêmes est plutôt la formation des prud'hommes en la matière. En effet, force de constater que les conseillers prud'hommes ne reçoivent qu'une formation rudimentaire en la matière. Voir aucune si les choses ne se passent pas très bien. Alors comment organiser une procédure de conciliation. Quand on lui est pas formés et comment on peut attendre une intervention des prud'hommes à laquelle on ne les formes guère. C'est pourquoi nous proposons par le biais de cet amendement de former les prud'hommes spécifiquement à la procédure de conciliation au moment de la formation initiale. Après leur élection. J'en viens aux dernières amendements sur l'article 8. L'amendement 236 qui consiste à accorder aux défenseurs syndicaux plus de temps pour l'exercice de leur mandat en période de renouvellement pour faciliter les candidatures. Les 4600 défenseurs syndicaux et sont essentiels pour le bon fonctionnement des conseils des prud'hommes le rôle 1er c'est bien évidemment d'assister les salariés tout au long de la procédure de représenter les salariés devant le conseil des prud'hommes et mais il et elle ont également une fonction d'ambassadrice ou d'ambassadeur pour le conseil des prud'hommes ils peuvent raconter leur expérience aux salariés motiver les gens pour pour candidater et nous avons besoin de ça parce que c'est aussi de plus de candidatures dont nous avons besoin si l'on veut combler le nombre de candidatures et donc remédier au au fonctionnement embouteillé des conseils des prud'hommes. Mais ce potentiel, il est aujourd'hui pas utiliser pleinement et un des freins, c'est que les défenseuse et défenseurs syndicaux bénéficient d'une autorisation d'absence qui est limité à 10h par mois et qui n'est pas. Flexible. Nous proposons simplement de l'augmenter de la doubler, je vous assure pas tout le temps mais uniquement lorsque nous sommes entend en période de renouvellement des conseils prud'homaux puisque nous considérons qu'à ce moment-là, hé bien il y a un travail important. Des défenseurs syndicaux pour pouvoir aller expliquer aux salariés. En quoi consiste le travail des prud'hommes. Pourquoi c'est intéressant. Pourquoi le faire et ce soit uniquement pendant cette période, mais nous considérons que ce serait peut-être un des. Une des procédures qui pourraient améliorer augmenter le nombre de candidatures, je vous remercie. Merci. Avis de la commission. Merci monsieur le président. Donc je vais aussi répondre sur l'ensemble des amendements donc le 1er. Of propose la possibilité d'être candidat aux fonctions de conseiller prud'hommes Sur son lieu de résidence en cas de télétravail de 30% de télétravail. Cet amendement qui étendrait a effectivement le vivier des candidats. Pour autant, il nous semble un peu imprécis quant à son impact a et crée une inégalité. Avec les salariés qui n'effectuent pas télétravail. Donc nous nous en remettons à l'avis du gouvernement. Nous comprenons le besoin d'élargir le vivier maintenant est-ce que c'est une. C'est quelque chose de réaliste et de réalisable. Le deuxième hein. Vous parlez. De restreindre en réalité puisque l'objectif. Affiché est de faire que les délégués syndicaux n'est plus à s'occuper. De l'activité de mandataire de listes mais du coup, l'amendement telle qu'il est rédigé ne ferait que restreindre les possibilités offertes aux délégués pour leur crédit d'heures et donc ça nous semble. Plutôt contreproductif. Mais. j'y reviendrai après puisque. On comprend que finalement vous allez doubler le nombre d'heures avec le dernier amendement. Ce qui réglerait ce sujet-là. Il n'existe pas de 40 d'd'article 40 ans qu'il s'agit d'augmenter les frais pour les entreprises. Pour autant, je pense que ça n'est pas forcément bienvenue et enfin l'article qui. Parle de la formation à la conciliation, effectivement le rapport d'Agnès Canayer de Nathalie Delattre. Faisait ressortir ce manque. C'était en 2019. Depuis, elles ont été entendues et cette formation aujourd'hui existe donc votre amendement est déjà satisfait retraite. Avis du gouvernement, sur les quatre un moment. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Vogel. L'un des objectifs de cette réforme. C'est une meilleure formation des conseillers prud'homaux. Nécessité d'améliorer la formation soulignait d'ailleurs de façon. Très explicite par les états généraux. Cela relève cependant davantage du réglementaire que de la loi. Et sur la. Le télétravail et le choix. Du domicile ou du lieu de travail. J'entends ce que ce que vous dites. Je souhaite que nous étudions davantage et que nous à Fignon davantage les chiffres. Le seuil de 30%. Je ai pas du tout certain qu'ils correspondent à la réalité. Il était si vous me permettez cette familiarité pris un peu au doigt mouillé. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable aux amendements que vous. Proposez madame la sénatrice. J'en déduis que la commission et donc sur le coup défavorable aussi aux 233 parce que c'était l'avis du gouvernement. Merci. Je vais mettre aux voix successivement ces quatre amendements qu'un avis défavorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour le 233. pour le 233. Même vote pour les 3 autres. Même vote, ils sont rejetés. Je mets aux voix l'article 8 qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Après l'article 8 l'amendement 248 Monsieur Mohamed sur. Conseil des prud'hommes réputée démissionnaire en raison du non-, respect de l'obligation de formation initiale. De faire une demande un relèvement d'incapacité. Le dispositif que nous vous proposons d'adopter partent du constat que certains conseillers prud'hommes dispose de motif légitime légitime justifiant le nom suivi de la formation initiale. Par ailleurs, nous proposons que le relèvement soit prononcée. Par arrêté et non par décret. Cet amendement prévoit un mécanisme similaire à celui des juges consulaires en matière de relèvement d'incapacité en cas de non respect de l'obligation de formation initiale. Nous y sommes donc favorables. et moi aussi, Monsieur le Président, parfait, je mets de vol 248 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Je mais on voit l'article 8 bis sans amendement qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Je vais avoir le 8 terre même chose qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Après le 8 terre le 213 Madame Billon. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à améliorer les modalités de mise en oeuvre de la parité au sein des conseils de prud'hommes il modifie 2 articles du code du travail l'Arctique elle 1441 19 qui encadrent le dépôt des candidatures lors du renouvellement général des 14.512 conseillers prud'homaux et l'article L. 1441 Tiret 29 qui encadrent le dépôt des candidatures prud'homale lors des opérations de désignation complémentaires lors du renouvellement général, les candidatures se présentent sur des listes qui doivent respecter une à l'alternance stricte des sexes lors des désignations complémentaire si un nombre équivalent de conseillers prud'hommes de chaque sexe siège déjà et qu'il reste au moins 2 sièges vacants la rédaction actuelle empêche le dépôt d'une seule candidature dans la mesure où cette candidature creuse l'écart entre les 2 sexes l'amendement revient donc sur ces difficultés algébriques en créant une dérogation permettant aux organisations qui se retrouveraient dans cette situation de pouvoir présenter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant à la moitié des sièges à pourvoir à un prêt dans le cas où le nombre de sièges attribués est un nombre impair des exemples m'ont été remontées du terrain, notamment le conseil des prud'hommes de Montmorency, où il y avait de candidatures féminines qui n'ont pas été déposée pour faute de candidats masculins ou par exemple à Bobigny, où il y avait 3 candidatures féminines sont d'ores et déjà identifiés mais aucun candidat à nouveau masculin donc où sont les hommes seuls, donc de candidatures féminines pourront être déposés. Donc l'idée c'est véritablement de pallier cet écueil et donc. Gagner en parité mais sans les difficultés je vous remercie. Merci madame la présidente. La vie de la rapporteure. Merci. Monsieur le Président. Alors madame la présidente. Effectivement c'est un assouplissement des règles de parité dans la mesure où 8% des juridictions prud'homales sont actuellement vacants fin de pneus des postes vacants sont vacants. La dérogation de cette parité semble bienvenue. Pour autant, nous pourrions faire un appel un peu poussé pour obtenir cette parité en n'ayant plus d'hommes. Mais écoutez puisque les femmes sont volontaires. Allons-y. Une douce pression comme d'habitude, madame la sénatrice. Non j'y suis totalement. Irrésistiblement favorable madame la sénatrice. Et. il y a évidemment le principe mais il y a aussi quelque chose de de pratico-, pratique qui m'intéresse beaucoup dans la mesure où 13% des sièges de conseillers sont vacants 1888 sièges. L'assouplissement vous proposez permettra de réduire cette vacances et permettra par conséquent à davantage de section conseil des prud'hommes de fonctionner.

Qui est contre adoptée je mets aux voix l'article 10 ans amendement qui est pour. Qui est contre Hadopi. Après l'article 10. Un amendement 258 Monsieur. Soleil. Oui, monsieur le président. Cet amendement vise à remplacer la référence aux conditions d'aptitude pour être assesseur du pôle social. Par une vérification que l'extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Ne comporte pas de mention incompatible avec l'exercice des fonctions. Nous souhaitons ainsi, comme pour le président ta maman. Aligner les conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux sur scène applicable aux conseillers prud'hommes. Merci. Alors ce serait un avis défavorable. Monsieur le Président parce que on comprend qu'il faille assouplir mais. Mais limitons-nous quand même dans l'assouplissement puisque cette amendement fait tomber de nombreuses incompatibilités et va au delà d'une simple simplification des conditions de candidature actuellement les conditions prévues sont notamment l'absence de condamnation pour. Crimes ou délits figurant au casier judiciaire numéro un que vous ne demanderiez plus la jouissance des droits politiques, civils, de la famille et de et de familles les personnes déclarées en état de faillite les fonctionnaires révoqués de leurs fonctions et tout cela n'y figurerait plus ça ne me paraît pas tout à fait.

Je suis favorable, parce qu'il simplifie la désignation des assesseurs des pôles sociaux en groupant les conditions de candidature au sein du seul code de l'organisation judiciaire et non plus par référence au Code de procédure. Pénale. Et supprimé la référence aux conditions d'aptitude pour être juré en matière pénale ne revient pas à ne pas exercer de contrôle. Puisque vous prévoyez un contrôle de l'absence de mention incompatible avec les fonctions d'assesseur au bulletin numéro 2 du casier. C'est d'ailleurs ce qui est prévu pour les autres juges non professionnels. Qui est contre. Il est rejeté. Le 259 encore Monsieur Mohamed soleil. Merci Monsieur le Président. Celui-ci. Vise à simplifier les modalités de prestation de serment des assesseurs des tribunaux pour enfants. Les assesseurs doivent actuellement prêté serment à chaque désignation qu'il s'agisse d'une première nomination ou d'un renouvellement. Ce dispositif est contraignant et coûteux pour les juridictions qui doivent organiser des audiences de prestation de serment pour toute désignation aussi, nous proposons de préciser dans le code de l'organisation judiciaire que seuls les assesseurs des tribunaux pour enfants qui n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein d'un tribunal pour enfants doivent prêter serment. Favorable, Monsieur le Président, cela nous semble une simplification bienvenue. S'il y avait du gouvernement même avis monsieur le président. Merci le 259 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Article 11, le 42. Madame de La Gontrie.

comme on veut, un thème très important me semble-t-il pour le bon fonctionnement de la justice qui est celui de ce qu'on appelle. Couramment l'équipe autour du juge. Inutile d'y revenir. Plus en détail tout le monde comprend. Ce que ce terme et. Précise. Et là cet article parle des notamment des attachés de justice. Et notre amendement vise à, à préciser un terme pourquoi dans l'équipe autour du juge il y a plusieurs types de professions médias les greffiers. Et donc il nous semble très important qu'il n'y pas de confusion entre la mission des greffiers et la mission des attachés de justice et donc nous souhaitons que le terme assistance. Qui est aujourd'hui prévue dans ce premier alinéa de de de de duel de 100 123 IV qui définit les attachés de justice ou les experts exactement leur mission qui soient parlait de soutien et non pas d'assistance parce que l'assistance. Cela relève des missions des greffiers. Je pense que si on veut que tout ça soit. Le plus fluide possible et le plus acceptée par tous, il faut que les missions de chacun soit très bien défini, c'est pourquoi nous proposons aux proposons le terme soutient et non pas le terme d'assistance concernant les attachés de justice. Moi je trouve que la différence entre effectivement le rôle des greffiers, on l'a dit. Largement dans nos débats et au monde. Discussion générale est fondamentale et on déplore que dans le cas de l'équipe autour du magistrat. La vision qui soit projeté aujourd'hui par le gouvernement et de ça de ce que nous espérions car nous pensons et nous le redisons, que les moyens supplémentaires sont extrêmement bienvenue et on s'en félicite néanmoins l'efficacité, la confiance ne sera restaurée que si véritablement il y a une réorganisation du travail à l'intérieur des juridictions et cette réorganisation, elle passe par une véritable équipe autour du magistrat qui associe. Les greffiers avec évidemment des attachés de justice et les assistants spécialisés. Mais nous pensons que votre proposition sémantique madame la sénatrice n'ajoute pas vraiment de la clarté au sujet donc nous sommes défavorables. je pense qu'effectivement Monsieur le Président Madame la sénatrice de la country c'est. C'est de la sémantique. Assistance soutient, bon ce qui m'importe. À ce stade c'est de rappeler que les greffiers sont les greffiers. Les attacher sont les attacher n'ont pas les mêmes fonctions. Non mais je ne vois pas pourquoi je vois pas pourquoi si on retient soutien. Ce serait plus clair. Les greffiers savent très bien qu'ils sont greffiers avec des fonctions de greffier qui sont essentiels et et les attacher son attaché vous changer un mot par un autre. Je ne vois pas trop ce que ça nous apporte en termes de plus-value. Je pense même que ça peut complexifier un peu les choses et je rappelle que la commission des lois a d'ores et déjà opéré une. Clarification très nette. Entre les missions qui sont confiées aux attachés de justice qui soutiendront les magistrats et ne pourront pas empiéter sur le fixe juridictionnelle des greffiers.

Qui est contre, il est rejeté. Peut être madame de La Gontrie. Si les trois concerne les attachés de justice pouvait présenter les trois et la Commission et le gouvernement donneront leur avis après ça prend des mesures pas vous le demander président c'est que du bonheur. Allez-y madame de La Gontrie. Alors le premier qui est donc le 43. le 43. De préciser. Les conditions dans lequel on peut être nommé attaché de justice en prévoyant hein. La nécessité d'un d'un diplôme. Formation juridique au moins égale à 5 années d'études supérieures. Aujourd'hui, tels que le projet de loi le propose. Les conditions permettant d'être nommé attaché de justice. Et donc notamment les conditions diplômes sont renvoyées un décret en Conseil d'État. Il nous semble que cela mérite d'être un petit peu plus précis et d'être. Clairement assez exigeants sur le le niveau de de recrutement et donc de limiter la portée du futur décret en Conseil d'État en prévoyant d'ores et déjà qu'il faut une formation juridique au moins égale à 5 années. Ça c'était le premier amendement le deuxième qui est le 44. Il s'agit des délégations de signatures les attachés de justice vont disposer au terme du projet de loi de délégation de signature dans un Champ extrêmement vaste. Notamment concernant les réquisitions toutes les réquisitions.

Donc on parle de de réquisition matériel il nous semble qu'il faut limiter le Champ d'application de la délégation de signature parce que c'est tout de même très lourd comme compétence et que les attachés de justice c'est très bien mais ils ne sont pas juge donc. Il nous semble nécessaire de de de les cantonner à un certain type de délégation.

Alors effectivement, nous pensons que ces attachés de justice sont une bonne chose, d'abord ça clarifie l'ensemble des. Des des des statuts qui existent aujourd'hui pour les sucres rapides les. Les contractuels de proximité et donc on va vers de la clarification qui est quand même le maître-mot de nos débats depuis plusieurs jours. Donc ça va, on y va, on va plutôt dans le bon sens avec le bémol que j'ai déjà émis que nous pensons que cette équipe autour du magistrat, elle doit être plus renforcée plus. mais concernant les diplômes des attachés de justice. Nous comprenons et nous nous associons madame la sénatrice de La Gontrie à votre recherche de compétences bien évidemment et d'exigence. De ses attachés du qui vont avoir des missions essentielles dans l'assistance du magistrat dans son office. Néanmoins, on pense que. La condition diplôme relève et doit rester du domaine réglementaire et que l'encadré en exigeant un niveau bac plus 5 c'est. Interdire de notamment mettre en place. Pourquoi pas de l'apprentissage pour avoir des attachés de justice qui sont en formation de master et qui vont à terme à voir leur ma ma soeur 5 mais qui se forme pendant qu'ils sont. Dans ces fonctions-là. Donc je trouve que c'est mettre trop de rigueur et s'est enfermé. Les attachés de justice dans. Un, un vivier trop restreint. Donc c'est un avis défavorable. Merci avait du gouvernement. Ah pardon, pardon, vous n'aviez pas donné sur le deuxième, allez-y. Ça c'est pour le 43 pour 44. Monsieur le le président c'est la suppression de la délégation de signatures en faveur des attachés de justice, notamment en matière de réquisition de données informatiques. Je trouve que si vous le retirer ses délégations vous priver toute la substance de leur action et ils n'auront plus ce rôle de véritable assistance et de soutien même au magistrat. Avis du gouvernement, monsieur le garde des Sceaux. monsieur le président, madame la sénatrice de la compris sur le. Le 43. Votre amendement aurait pour effet. De supprimer la possibilité pour les titulaires d'un diplôme de doctorat en droit d'accéder directement à la fonction d'attaché de justice. Non, je ne puis naturellement qu'être défavorable à cet amendement. Sur le 44. C'est une délégation qui est une délégation technique. Oui et le magistrat reste le Capitaine de cette équipe. équipe. S'agit pas du tout, de permettre, il ne faut pas. Qu'il y ait d'ambiguïté dans les dans les esprits et de troubles s'agit pas du tout, de permettre un attaché de justice, de signer un jugement parfaitement compris, ni même d'ailleurs ni même d'ailleurs des réquisitions tels qu'on les entend classiquement prise par le procureur de la République. Non c'est pas ça. Mais. Vous ne voulez pas de l'assistance. Mais vous voulez du soutien mais vous enlevez une part de ce soutien, je veux bien aller vers vers ce mot parce que pour moi ils sont équivalents, mais ce n'est pas conforme à ce que nous souhaitons faire je veux dire un seul mot là-dessus, pardon monsieur le Président, je vais aller vite. Mais quand on les a mis en place ces contractuels qui ne s'appelait pas attaché de justice. Ils s'appelleront attaché de justice quand le texte sera voté. On nous a regardé avec beaucoup de circonspection. Et puis un an plus tard, les chefs de juridiction m'ont demandé qu'il soit pérennisé. C'est la raison pour laquelle nous les pérennisons nous les CD. Ils ont et nous leur demandons de recevoir une formation, et de prêter serment pour qu'ils soient mieux intégré dans cette équipe nouvelle qui va se former et qui va aider nos magistrats. Nos greffier qui en ont bien besoin notamment aller plus vite parce qu'un juriste assistant à côté d'un magistrat, c'est 2 fois moins de temps pour rédiger une décision et j'indique que ces contractuels ancienne mouture ont permis une réduction extrêmement importante des stocks endémique d'affaires civiles, qui font que la justice est si lente. Merci je vais mettre aux voix d'abord le 43 plus de 44 avec 2 avis défavorable qui est pour le 43. Contre. Rejetée même vote pour le 44 même vote. Le 272 du gouvernement, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le président. Dans le cas de l'assistance ou du soutien. Je souhaite pour être plus efficace encore que l'on permette la levée du secret fiscal à l'égard des assistants spécialisés. Invité de la commission. C'est un avis favorable parce que ça correspond à une recommandation du rapport de notre collègue Jean-François Husson, sur la lutte contre la fraude fiscale. Ciao bouleversé. Je mais on voit le 272 du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Il est adopté, je mets aux voix l'article 11 qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. À l'article 12 l'. 280. De la commission des lois. Merci, monsieur le Président, donc c'est un amendement qui apporte une précision concernant la création d'un conseil de juridiction auprès de la Cour de cassation. De manière à ce qu'il y ait une représentation conjointe du procureur. Général à côté du 1er président. Personnellement. Favorable, monsieur le président. Merci je mais aux voix l'amendement de la commission avec un avis favorable du gouvernement le 280 inquiet pour. Qui est contre, il est adopté. Je mais aux voix. L'article 12 qui est. Pour. Qui est contre. Il est adopté. Après l'article 12, le 260 Monsieur Mohamed soleil. Oui, monsieur le président, il s'agit d'un amendement rédactionnel. Qui vise à remplacer une référence lié à la désignation des tribunaux judiciaires spécialement compétents pour connaître des litiges liés à l'ouverture l'abonnement et l'utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Article 13. J'ai d'abord 2 amendements en discussion commune le 281 de la commission. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement. Été rédigé en concertation avec le Conseil national des barreaux et il concerne la procédure disciplinaire des avocats. Alors ils visent à à faciliter la désignation de rapporteurs en phase d'instruction et de membres des conseils de discipline. Et d'assesseurs dans les formations de jugement en Cour d'appel.

Qui est contre. Il est adopté le. 83 tombe et par conséquent, nous passons à 2 autres amendements en discussion commune le 282 de la commission, madame Canayer. Oui, merci Monsieur le Président. C'est la cet amendement vise à créer une procédure disciplinaire simplifiée du plaider coupable pour les avocats. Merci. Toujours en discussion commune le 84. Monsieur anglaise monsieur Charon. Il est défendu. Il a défendu avis de la commission sur le 84. Il est très proche d'une autre donc demande de retrait au profit de l'amendement de la commission. Merci avait du gouvernement sur les deux. Même avis. Monsieur le Président, au pluriel. Il est retiré donc je mets aux voix directement le 282 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement qui. Pour. Il est adopté. Le suivant et retiré le mais aux voix l'article 13 qui. Pour. Qui est contre. L'article 13 est adopté à l'article 14. Juin 147, monsieur Bena Roche. Oui il est bien à moi. Monsieur le président. Une fois de plus, bien entendu. Nous saluons le fait que ce projet de loi développe des moyens financiers pour la justice souhaite régler les problèmes de manque de personnel et faire gagner en attractivité les professions qui pâtissent de ce sous-effectif nous saluons cet effort. Mais si la création d'emplois et sur les tables, les modalités de recrutement imaginer. Dans cet article par le gouvernement nous paraissent plus que contestable. La mise en oeuvre de de surveillants pénitentiaires adjoints contractuels devant pallier le capital insuffisant. Dans des services pénitentiaires nous Jacquiet c'est surveillants Adjoua seront peu formés. Sera amené à effectuer des missions de sécurité sur les détenus. De participation à l'individualisation de leur peine, ainsi qu'à leur réinsertion, ce qui nécessite une formation importante et aussi une date du Mans formés à la relation avec les personnes détenues. Dans un 2ème temps. Le choix de la contractualisation de l'emploi est regrettable parce qu'il traduit à statut précaire est stable peu attractif qui ne fait qu'apporter des réponses de court terme, on l'a bien vu puisque vous transformer un certain nombre de contrats dans d'autres domaines. Qui étaient des contractualisation voulait supprimer pour en faire des des des contrats. Fermes. Nous inquiétant donc de ce potentiel glissement vers la côte. Contractualisation en tout cas du personnel pénitentiaire. En plus dans cet article 14. Vous pérenniser l'utilisation des caméras piétonne dans l'expérimentation au cours avait pour but de prévenir les violences et d'amis il y aurait la sécurité en détention. La possibilité de transmission en temps réel des images à poste de commandement pose problème dès lors que l'accès Direct à ces images par les personnes concernées n'est pas prévu. Par ailleurs le clean. A révélé que ce dispositif n'a ni amélioré les conditions de travail des agents de l'administration pénitentiaire ni eu un impact positif sur des résolutions des incidents. Nous demandons donc la poursuite de l'expérimentation pour apporter de meilleures garanties au dispositif merci. Il avait de la commission. Ce sera un avis défavorable. Monsieur le Président, puisque notre collègue ben arrange nous propose de supprimer cet article sur les surveillants adjoints contractuels. C'est vrai qu'au départ, nous étions aussi un peu dubitatif. À la Commission doit parce qu'on comprenait pas très bien l'enjeu. Et quand tous deux a expliqué que c'était des emplois-, tremplin pour favoriser le recrutement. Des surveillants alors qu'aujourd'hui il y a un vrai problème d'accès à ces emplois. Nous en avons compris la finalité. Moi je travaille beaucoup dans les missions locales à côté de l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et on voit aujourd'hui qu'il y a un ensemble d'offres d'emplois dans la fonction publique d'État et des collectivités territoriales qui manque d'attractivité qui ne sont pas connues et pour lesquelles les jeunes ont du mal à s'orienter. Et je trouve que cette idée est donc une très bonne idée. Elle va permettre. D'intégrer des jeunes et de les sensibiliser à ces emplois. Qui sont aujourd'hui peu attractif

Les détenus. Il faudra bien qu'on a sur leur garde. On a bougé les catégories. Vous savez, c'est une revendication qui a plus de 20 ans. Tout ça est une question d'attractivité. Ce que nous mettons en place. Va permettre justement de régler ces questions, je suis évidemment défavorable à votre. Amendement monsieur le sénateur, ben.

vote. Sur quelles bases d'articles. Que sur un vote c'est purée. Article 42, alinéa 11 du règlement, Monsieur le Président, nous souhaiterions demander un vote par division de cet article qui traite dans un 1er temps, des surveillants. Adjoint entre 18 et 30 ans. Auxquels nous ne sommes pas favorables et qui traite dans une 2ème partie des caméras individuelles. Donc c'est pour cela que je me permets de demander un vote par division afin que nous puissions nous exprimer sur les deux sujets de manière distincte. Madame de La Gontrie. Le vote sur l'article n'est qu'à la fin et nous sommes obligés de faire les votes d'abord par amendement. Donc nous verrons. D'abord, après le 147 si oui ou non l'Assemblée d'accord pour procéder au vote par division. Sur le 147 donc je reviens. Qui est l'amendement de suppression, je le rappelle de l'article avec 2 avis défavorable qui est pour.

Wim ce président un amendement rédactionnel qui vise à renvoyer la définition de conditions de formation des survient adjoint à un arrêté et non à un décret en Conseil d'État. Donc nous demandons de la souplesse. Merci. Avis de la commission. Sagesse. Avis du gouvernement. Favorable. Très bien. Donc sur le 223. Sagesse de la commission favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Le 61. Madame de La Gontrie. monsieur le président je je je pense je n'aurai pas besoin à nouveau tout à l'heure au moment du vote de l'article de redemander le vote par divisions. On est d'accord. 2ème set 2ème partie donc de de l'article. 14 très de. L'instauration de caméras individuelles dont seraient dotés les surveillants et qui permettrait ainsi en cas de d'incidents. d'avoir toute une série d'éléments qui permettraient d'en connaître. La genèse. Nous y reviendrons longuement il y a de nombreux amendements et beaucoup de modalités cet amendement prévoit que. Ces caméras ne peuvent pas être. Activé au moment d'une visite médicale afin que le secret médical soit préservé et donc il faut que ce soit prévu expressément, me semble-t-il, voilà l'objet de cet amendement. Ce sera un avis défavorable. Parce que la formulation de votre amendement est beaucoup trop large. Il est normal qu'il puisse y avoir des caméras dans. Les transfèrements dans les salles d'attente et d'autres, d'une part et d'autre part durant la consultation c'est impossible puisque c'est déjà protégés par le secret médical. gouvernement. Oui oui oui. Monsieur le président. Même avis je mets aux voix le 61 avec, ah pardon madame de La Gontrie. Merci président. Moi je veux bien toutes les circonvolutions de la rapporteure. Mais ce texte a été écrit plusieurs fois, je note qu'elle ne propose pas de rédaction alternative. Lorsqu'on parle de visite médicale, on sait très exactement. Alors si vous le souhaitez, on peut parler de l'examen médical. Mais on voit quand même de quoi on parle, c'est-à-dire qu'un détenu est en train d'être examiné par un médecin. Je considère qu'il n'est pas acceptable de permettre que cet examen médical soit filmé. Donc vous ne le voulait pas, dont acte, mais en tout cas, ce ne sont pas vos explications qui permettent d'être convaincant. Madame la rapporteur. Merci monsieur le président. Mais vos explications, madame la sénatrice de La Gontrie, ne le sont pas plus puisque c'est d'ores et déjà protégés pendant un examen médical pendant pendant une consultation médicale ses protégés par le secret médical, De de de de de prise de vue et ça ne peut pas être filmé donc parce qu'on va pas rajouter du droit au droit, quand c'est déjà prévue par le droit, je ne vois pas l'intérêt de rapport de de remettre des dispositions qui sont en plus trop vagues, puisque vous englober tous.

donc votre amendement, il est trop globales. Il est trop large, d'une part et d'autre part je redis que pendant la consultation c'est déjà protégés par le secret médical. Merci

C'était le 196 Madame du birmane. Oui merci à Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux à travers cet amendement, nous souhaitons que les personnes utilisant des caméras individuelles doivent justifier de raisons matérielles, concrètes, les ayant empêchés d'informer les personnes enregistrées. Cela permettra de limiter les restrictions d'information situation des contraintes matérielles réelles et objectives empêchent la communication et d'éviter de laisser place à de justifications vagues ou abusive. Cette clarification nous semble nécessaire pour garantir la transparence, la responsabilité de l'utilisation de tels dispositifs. pardon. Nous comprenons pas très bien la portée de votre amendement notamment cette notion de circonstances matérielles qui nous paraissent un peu flous on pense qu'aujourd'hui le dispositif prévu est. Satisfaisant et que il n'y a pas besoin de, de préciser les notions. Donc c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement. Défavorable. Monsieur le président. Merci je mais aux voix le 196 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Le 45. Madame de La Gontrie. Merci monsieur le président je je regrette que. L'ensemble de ce dispositif soit appréhendé avec un peu de légèreté. Parce que je pense qu'il est important et utile. Il est utile pour les surveillants pénitentiaires. Il est utile pour les détenus et cela peut éviter beaucoup de suspicion de contentieux, ça peut éviter permettent d'éclairer en cas de procédure disciplinaire donc. Nous y sommes. Globalement favorable, dès lors que cette encadré l'article. 11. Dit déjà beaucoup de choses en terme d'encadrement. Mais la question est de savoir à quel moment l'information est délivré de cette. De de cette possibilité de de filmer. Donc c'est pour cela que. Nous demandons qu'il soit prévu qu'elle soit au plus tard au terme de l'intervention. Il faut que les personnes sachent qu'elles sont filmés. Avis de la commission. Ce sera un avis. Défavorable. Parce que on sait effectivement la place des caméras individuelles est importante, elle était attendue, elle est attendue notamment par le personnel des établissements et donc c'est un sujet, on le sait bien. D'importance. Néanmoins. C'est pas la peine d'alourdir non plus le dispositif parce qu'il faut aussi que l'utilisation. Des images. Tout dans, dans le cadre du respect évidemment des droits de la défense mais que l'utilisation des images puisse être réalisée de manière effective effective et efficace et donc nous pensons que les modalités d'information des personnes sont d'ores et déjà prévue par l'article 14 qui dispose que l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent rajouter des délais ne nous paraît pas être une disposition qui améliorera significativement le dispositif des caméras.

le 197 madame vulgairement. Oui merci à monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, il me semble important de pouvoir introduire une disposition spécifique visant à informer les mineurs incarcérés, qui est un public particulièrement vulnérable de l'utilisation des caméras individuelles par les agents pénitentiaires. Nous considérons en effet qu'il est essentiel de garantir que les mineurs détenus soient informés de manière claire adapté. Concernant la possibilité d'être enregistrées par les caméras individuelles. Cet amendement vise donc à protéger leurs droits et à prendre en compte leur situation spécifique. Et la commission. Défavorable. les instructions qui sont données aux personnels pénitentiaires. Sont les mêmes et elle consiste à ce que l'information soit délivré dès que possible et au plus tard au terme de l'intervention, ce qui est d'ailleurs conforme aux recommandations de la CNIL défavorable. Merci je Metz de voix le 197 avec 2 avis défavorable qui est pour.

Qui est contre. Adopté. 3 amendements en discussion commune le 198 madame Cukierman. Oui, merci monsieur le président, Monsieur K garde des Sceaux. Un autre amendement a pour objectif d'établir le droit pour le détenu ou son avocat de pouvoir accéder directement aux enregistrements qui le concerne, réalisée à l'aide des caméras individuelles par les agents pénitentiaires. Actuellement, les agents ont un accès Direct aux images enregistrées tandis que le détenu, son avocat ou seulement un accès Direct par le biais de la CNIL. Cette disparité d'accès limite les droits de la défense dans certains cas, afin de garantir l'effectivité des droits de la défense. Nous considérons qu'il est primordial que le détenu ou son avocat puisse accéder directement aux images enregistrées par les caméras individuelles. Cette disposition permettrait ainsi de renforcer, comme je l'ai dit précédemment, la transparence, l'équité du système pénal en donnant aux parties concernées, la possibilité d'examiner les preuves à charge ou à décharge de manière directe et sans délai excessif. Ah c'est en discussion commune pardon le alors 2 amendements identiques le IV. D'abord monsieur Fischler. Oui. Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, c'est une forme d'amendement de repli puisque il vise à prévoir l'accès par l'avocat de la personne détenue des enregistrements qui la concerne, alors que les agents qui filme auront un accès Direct aux images. Cette possibilité est actuellement limité pour le détenu et son avocat. A un accès indirect via la CNIL afin que les droits de la défense soit effectif, il nous apparaît nécessaire que l'avocat puisse accéder directement aux images. Merci identique monsieur Bena Roche le 136. Oui donc je vais pas être très or puisqu'ils auraient été parfaitement défendu par mes deux collègues auparavant je rajouterais juste quand même que cet amendement est issu des travaux du Conseil national des barreaux. Merci. Avis de la commission sur les trois amendements. Merci monsieur le président, alors. Ce sera un avis défavorable sur ces trois amendements. Parce qu'aujourd'hui on pense qu'il y a une procédure déjà suffisamment solide sous réserve de suffisamment solide en matière d'accès. Aux images, notamment via la CNIL sachant que le directeur de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer si nécessaire mais devra justifier cette opposition. Sous réserve de. Sous réserve que le décret. D'application soit adoptée parce qu'aujourd'hui il reste encore. À encadrer et c'est renvoyé un décret qui n'a toujours pas été adopté donc avis défavorable pour les trois. Merci avait du gouvernement triplement défavorable triplement défavorable. Très bien. Eh bien je vais mettre aux voix d'abord le 198 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Rejeté puis les 2 amendements identiques, le 4 et le 136 quai pour. Qui est contre. Rejeté. Je passe. 56. Madame de La Gontrie. Merci monsieur le président. Lorsque nous avons eu ce débat en commission. Il avait déjà été indiqué que libre aux détenus de s'adresser à la CNIL. On voit bien qu'on n'est absolument pas dans la même temporalité. Et donc l'amendement que nous proposons prévoit expressément le cas de la procédure disciplinaire. C'est-à-dire que si une procédure et mise en oeuvre. À l'encontre d'un détenu voir avant qu'on a surveillant, mais en l'occurrence d'un détenu. comment se passe le le la récolte des éléments de l'infraction éventuelle si on ne peut pas avoir accès aux images. Donc on a un problème de droit de la défense. On a un problème de contradictoire et donc cet amendement est au fond une sorte de repli par rapport à ceux qui ont présenté par les collègues précédemment et qui prévoit expressément la communication possible si cela est demandé. En cas de procédure disciplinaire.

qui prévoit la procédure disciplinaire et qui prévoit que c'est un décret qui détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à disposition et celle dans lequel l'avocat ou la personne intéressée si elle n'est pas assisté d'un avocat peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. C'est ce décret qui doit fixer cette procédure. Je pense qu'il n'est pas utile de la mettre dans la loi, il faut surtout demander à monsieur le ministre que ses services lui propose rapidement l'adoption de ce ce ce décret qui permettra d'encadrer plus clairement l'accès notamment aux images. Des caméras individuelles votre amendement est d'autant plus. D'acceptable que. Il fait il supprime toute la possibilité pour le directeur de l'établissement de s'opposer à. La transmission des images et à l'obligation de l'administration de justifier auprès de la CNIL, son refus d'accès à ces images, qui sont pour nous des garanties importantes donc avis défavorable. Avis du Gouvernement. Défavorable. Le décret sera pris très rapidement.

Oui mais c'est le président cet amendement vise à inscrire dans le code pénitentiaire, la procédure alternative aux poursuites disciplinaires. Cette procédure permet d'apporter une réponse rapide à des incidents de moindre gravité mais fréquents en détention. Elle présente également l'Avantage de privilégier des mesures de réparation et de médiation. L'encadrement juridique de cette procédure permettra d'harmonisation et la sécurisation juridique des initiatives locales, déjà en place. Merci. Avis de la commission. Ce sera un avis favorable cette cette mesure nous paraît. Intéressante. Pour notamment le pacifier j'imagine les relations au sein des établissements pénitentiaires, peut être qu'elle a besoin d'être étudié plus de manière plus approfondie mais nous donnons un avis favorable. Mercier avait du gouvernement. Je trouve que c'est un excellent amendement. Mais vraiment. Et et ça va dans le sens de la médiation. que je porte en matière civile et que je veux porter également en matière pénale, c'est à la fois de la fermeté mais c'est aussi de la responsabilisation. Du du détenu. Ça me paraît aller dans le bon sens. Je suis vraiment très favorable à cet amendement.

Il est adopté. Je vais passer l'ensemble du vote à la demande de madame de La Gontrie, d'abord, avis de la commission là-dessus puisque. L'article 42 alinéa 11 prévoit éventuellement que la commission demande la commission demande C'est un avis défavorable. Monsieur le président. Un avis défavorable. Monsieur le prix. Alors pardon pour la commission je prends sur moi de faire quand même ce vote par division puisque le président décide et c'est bien ainsi. Parce que ça ne change pas grand chose, si madame de La Gontrie en est d'accord, je propose un vote des alinéas hein puis des alinéas 9 à 21, section 3 puis La Linea 22 et ensuite évidemment un vote sur l'ensemble donc 3 votes divisionnaire puis un vote d'ensemble. Est ce que madame de La Gontrie. Cela pourrait vous convenir. Cela vous convient. Il en est ainsi décidé je mets donc aux voix les alinéas 1 à 8 de l'article 14 qui est pour.

Qui est contre. Hadopi. Merci. Je passe. À l'article 15. Avec 3 amendements identiques d'abord le 46. Madame de La Gontrie. Merci monsieur le président. Et merci de du vote par division qui vient d'être opéré. Cet article. Je l'appelle un petit peu un petit peu l'article.

Et donc. Ici nous avons. Alors le garde des Sceaux tout à l'heure, je suis sûr nous dira avec. Beaucoup de conviction dans la voie qu'il s'agit de plus de souplesse et cetera et cetera mais on Un mécanisme qui se met en place qui a vocation à permettre. Des transferts de compétences sur un certain nombre de sujets qui relèvent tous des libertés. Et qui ne soit pas forcément exercée par le juge des libertés et donc on voit bien que il y a vocation ainsi à compenser de de de de magistrats dans un certain nombre de domaines pour le confier à d'autres. Ce qui est préoccupant, c'est que bah d'abord la pratique des libertés, c'est quelque chose de, de très particulier, c'est une compétence spécifique et que donc ça nous semble dénaturé. La mission des des JLD en la rendant incomplète et c'est pour cela que nous souhaitons la suppression de cet article. Merci monsieur Bénard Roche le 137. Oui, monsieur le président. Le le mouvement depuis de nombreuses années consiste. À ajouter de nouvelles missions. À celle du du du juge. Des libertés et des tuteurs sur ce soir. Je crois qu'il y ait une réelle cohérence. Une vision d'ensemble d'ailleurs des missions qui lui sont. Donc ça fait une charge augmenter avec un nombre de juges en sous-. Effectif. Ce qui crée des conditions de travail particulièrement difficile, ce qui explique d'ailleurs que ce nombre de juges sur sous-effectifs qui sont liés à la fonction. Les horaires sont décalés, les audiences sont tardive. Il y a des permanences de nuit et le week-end, il faut le savoir si vous d'avoir n'importe quel GLD vous le dira. Il est de permanence. La nuit et le week-end. En fonction du nombre de GLD quand il y en a que deux et sur en permanence une fois sur deux. Leur mission première de contrôle des libertés des personnes sous main de justice de retenue de détenus ou de les enfermer sont donc de plus en plus difficile à exercer. Donc nous regrettons cette surcharge de ces juges spécialisés mais au lieu de recentrer. Leurs missions, sur les points sur lesquels ils sont spécialisés. Ou bien de multiplier les recrutements nécessaires sur ces postes. Ce qui est difficile effectivement vu les conditions actuelles le gouvernance. Le gouvernement en fait propose de les dessaisir de leurs prérogatives en ce qui concerne le droit des étrangers et les prolongations des soins sans consentement. je connais les problèmes liés à ces pics d'activité. J'étais sur place lors de l'épisode Océan Viking. Bon. Mais l'ensemble des acteurs du terrain. L'ensemble et j'en ai rencontré plusieurs et encore dernièrement la semaine dernière à Grasse nous confirme que les dispositions du code de l'organisation judiciaire permettent déjà l'arrivée et le soutien un appui ponctuel d'autres juridictions. Le dessaisissement spécifique sur ces missions-là nous paraît aberrant parce qu'il part d'un constat juste de surcharge de travail. Et il il répond de manière purement gestionnaire et à côté de la plaque, oserais-je dire, Monsieur le Ministre, en retirant les missions qui sont au coeur de l'Office de ce JLD en les confiant à un juge non spécialisés. Je voudrais une explication de vote pour terminer. Merci monsieur le président. Donc les amendements proposés là propose de supprimer le transfert des fonctions civiles du juge des libertés et de la détention. Un magistrat du siège. Tout d'abord. Nous devons partager ce constat que l'accroissement continu d'émission du JLD et peu contestable. L'augmentation de leur charge de travail. Difficilement soutenable. J'entends bien, on pourrait embaucher plus, sauf que. Aujourd'hui, 16% de taux de vacance sur ce type de poste. Et le rapport des états généraux de la justice y voit une conséquence directe de la croissance du contentieux civil c'est donc bien parce que il y a trop de contentieux civil qu'il y a moins de JLD donc rajouter. Des postes qui ne seront pas remplies. Alors qu'on n'aura pas retiré ce qui les fait fuir ne réglera pas le le sujet. Par ailleurs, je rappelle que le JLD. À l'origine était conçu comme un tiers impartial disposant de suffisamment d'autorité pour déjuger d'un de ses pairs au cours d'une procédure. Or ce besoin n'existe pas dans les matières purement administrative qui sont celles sur lesquelles on transfère justement l'émission du JLD, un juge du siège que sont le droit des étrangers et l'hospitalisation sous contrainte. Donc on a plus besoin d'avoir cette spécialisation du JLD justement sur ces matières civiles et c'est pourquoi ceux-là peut être transféré à un juge du siège. Je continue sur le fait que du coup c'est ça ne ça ne effectivement pas de problème pour. Pour le Conseil d'État, puisque effectivement c'est les magistrats du siège hein dans leur ensemble sont les garants de la liberté individuelle et pas les seuls JLD. conjure moi je conclus en disant que rien n'interdira que le JLD continuent à assumer ses missions là où ce sera possible, mais ça donne une souplesse nécessaire. Merci à du gouvernement. Si Monsieur le Président, madame la sénatrice de La Gontrie pas Shadoks pas de sapeur Camembert pas Djiby tout simplement des choses. Pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous disent les magistrats. Ils nous disent. Vous savez, on a besoin que vous nous fassiez confiance sur le terrain. Aujourd'hui pour avoir une armoire métallique, il faut passer par la centrale magistrat dit Stop arrêtez faut déconcentrer n'importe. Laissez-moi terminer. Madame la sénatrice. Souffrez que je vous réponde. souffrait encore un peu, je vais être bref, moi vous m'interrompez moi vous souffrirai. Relation RH pareil et tout doit remonter par la centrale les JLD. Qu'est-ce qu'ils disent, ils disent, on a un contentieux qui est devenu de plus en plus important d'où l'idée. De faire en sorte que sur place les chefs de juridiction voit avec leurs JLD et qu'on puisse les décharger d'une partie du contentieux. Au profit d'un juge. De l'Ordre judiciaire, ça va de soi, appartenant au au même tribunal judiciaire étant lui aussi garant de la liberté individuelle, de par les termes de notre constitution. Pas plus compliqué que ça. Il y a des JLD qui disent on veut tout le contentieux, il y a des GLD qui disent on en a un peu trop, c'est pas à moi de régler ça de façon caporaliste. Pas de fantasmes. Pas de mauvaise idée. C'est tout simplement pratico-pratique donc les JLD qui renvoie à leurs chefs de juridiction pour dire j'aimerais bien un petit coup de main ben chefs de juridiction pourrait y être sensibles. Les JLD qui liront veut tout conserver, et ça va très bien comme ça conserveront tout voilà c'est simple. Le projet de loi que je porte, il a pour but de simplifier les choses.

c'est le contentieux en droit des étrangers, celui concernant le code de la santé publique, dont c'est la complexité et dont on sait qu'il nécessite plus que d'autres peut-être surtout celui sur le droit des étrangers, on est bien placé tous ici pour le savoir. L'examen d'un juge spécialisé. Ce sont des litiges qui sont de nature politique, on peut le dire. Alors que c'est c'est c'est de litige là. Et la délégation dans ce cas-là elle est source d'inquiétude forcément en plus de sa période. Permettez-moi de vous dire que ça met pas en situation facile non plus. Le le le juge qui va décider le le le président qui va décider. Parce que. C'est lui qui va avoir le pouvoir. Le président de juridiction de désigner, via une ordonnance de roulement, les magistrats qui se verront attribuer les fonctions du JLD. Donc il y a quand même quelque part là aussi. Près d'inquiétude et en plus j'ai pas rencontré à JLD qui m'a dit qu'il voulait être dessaisi de ce litige et donc même quand ils ont trop de travail parce qu'on leur a donné plus vous bien entendu. On leur donne de plus en plus enfin moi j'en ai pas rencontré, je ne sais pas dit que vous en avez pas rencontrée. Je n'en ai pas rencontré. Voilà et donc monsieur le garde des Sceaux. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait en surcharge de travail un certain nombre de fonctions et après on dit ben on va vous permettent de vous en enlever alors la relève ce sur lequel ils sont les plus compétents. Je ne voit pas la logique du raisonnement. Simplement pour dire que le week-end, ça se passe déjà comme ça. Il y a des magistrats qui sont pas JLD qui prennent la place de JLD ça tourne dans les juridictions puis ça marche. Voilà, ça c'est l'avantage de venir de la société civile puis de connaître un peu l'écosystème. Merci monsieur Monsieur le président. Merci monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues. Tout ça n'est pas anodin. Parce que vous nous dites ce monsieur le garde des Sceaux que ces pratico-pratique. Alors vous êtes devenu d'un pragmatisme intégral. Les JLD. Il faut un travail mais les autres juges du ressort peuvent également faire le même travail. Pourtant j'avais compris qu'il y avait une spécialisation et que celle-ci était particulièrement importante s'agissant des personnes venues des étrangers s'agissant des demandeurs d'asile. Vous savez que c'est un sujet très sensible par rapport auquel nous sommes dans un brouillard très grand. Puisque. Nous ne savons pas comment va se passer la future législation sur les immigrés. Et sur le droit d'asile. Nous avons entendu ce qu'a dit madame, la Première ministre. Nous avons entendu ce que dit monsieur le président de la République. Nous avons même entendu ce que dit le groupe LR. Ou un certain nombre de représentants du groupe LR ici représentés largement. ça nous avons vu un certain nombre de changements considérables dans la logique qui est celle du groupe LR par rapport à son histoire et même à son histoire récente. Donc dans ce contexte particulier qu'on ne peut pas ignorer. Il est légitime de se poser les questions. Ce que nous posons sur l'aspect purement pratico-pratique de ce qui est ici présenté et qui change quand même beaucoup d'articles du code du Ceseda et cela n'est pas anodin.

Qui est contre adopté. Je me vois l'article 16 qui est pour. Qui est contre adopté. À l'article 17 2 amendements identiques. Le 47. Madame de La Gontrie. Merci Monsieur le Président, nous abordons un nouveau thème. Parce que ce projet de loi est très varié. Qui est la question des saisies rémunération. Je pense que beaucoup de nos collègues ont été interpellés sur ce sujet,

Donc. Il faut savoir qu'évidemment ce ce ce le contentieux de rémunération est un contentieux à la fois banales et extrêmement. Volumineux c'est un contentieux de masse et donc on voit bien l'idée qui a été de se dire on va décharger les magistrats et confiée au. Haut commissaire de justice mais cela pose plusieurs problèmes, d'abord ça ne va pas aller plus vite. Puisque la procédure qui a été. Retenue ressemble comme une soeur jumelle à celle qui a été prévu précédemment avec un magistrat mais surtout. Cela va renchérir le coût pour les personnes concernées. Pourquoi vous le savez très bien lorsque il y a une mesure d'exécution. Il y a ensuite la facture arrive. Et la facture, c'est la première, c'est les frais du commissaire de justice qui vont donc être évidemment plus important puisqu'ils vont remplir une fonction qui ne remplissaient pas auparavant. Ensuite les intérêts ensuite l'ex-capitale et donc nous sommes des magistrats qui nous ont. Alertés lors de nos auditions avec la commission un renchérissement très important donc on revient. Non pas au sapeur Camembert mais en tout cas on se on se défausse en transférant commissaire de justice au détriment des créanciers et donc des débiteurs pardon et donc évidemment. C'est très préoccupant, car il s'agit toujours de personnes avec peu de moyens. Et qui sont de ce fait pendant longtemps des mois en grande difficulté. très belle présentation de de Marie-. Pierre de La Gontrie. Je je dirai 2 choses, d'abord je rappellerai ce que dit le Conseil d'État. Il s'est interrogé, ouvrez les guillemets sur les effets tant sociaux sur une population souvent vulnérables qu'une dérive même modique des coûts maintiendrait dans l'endettement. Qui économique privant les créanciers. D'une part peut être plus importante de ce qui leur revient donc c'est du perdant-perdant. En fait dans la réalité. De plus. On va dire même dans une cohérence de ce de ce projet de loi et c'est ce qui aujourd'hui nous rend dubitatif sur notre vote global. Monsieur le garde des Sceaux. En supprime un passage devant le juge qui nécessite actuellement une tentative de conciliation entre les parties. Vous avez vous-même souligné, il y a quelques minutes. L'intérêt d'un amendement de 2. Thani Mohamed Soilihi qui remettait de la médiation et de la conciliation là vous en enlever alors que vous êtes fixé en tant que gouvernement comme objectif inscrit dans le rapport annexé du même projet de loi. Qu'il fallait développer les conciliation et la médiation dans les prochaines années. Donc, ni du côté efficacité ni du côté cohérence politique. Je ne vois

Il ne s'agit pas d'un créancier qui va aller voir l'huissier de justice. Au bout de sa rue en disant monsieur machin me doit de l'argent ces c'est lui son salaire pour me rembourser. Ça n'est pas ça, puisqu'il faut qu'il y ait initialement un titre exécutoire, c'est-à-dire pour tous les créanciers privés être déjà passé par le juge qui aura donc admis que cette créance existe et qu'il faut la recouvrer

En insistant effectivement sur le fait que le commissaire de justice. Outre le fait de vérifier que cette créance est effectivement du alors là je ne pense pas à la partie juge mais la partie administration publique qui peut effectivement se tromper. Mais. Outre cela, on lui a demandé de d'organiser. Initialement, le la la négociation une phase amiable de recherche d'un accord entre le créancier et le débiteur. Avant d'en arriver à cette saisie sur rémunération dont je précise, vous dites que ce sont des gens qui ont de faibles revenus, pas toujours. Un mauvais payeur peut être tout à fait riche hein et ça. N'exclut absolument pas des personnes qui ont déjà tous un salaire par définition puisque c'est une saisie sur rémunération et donc ils ne sont pas toujours. Un sujet qui Par ailleurs, nous avons aussi souhaité simplifier la saisine du juge de l'exécution en cas de contestation malgré tout. Et ce serait c'est par simple requête je regarde. Notre collègue Mohamed Soilihi puisque je sais qu'il veut retirer cette mesure. Ça nous paraît assez simple parce que pour le coup le justiciable. Ça lui permet de juste envoyé un courrier sans être obligé lui-même de saisir un huissier. Et enfin nous

Le rôle du rapporteur. C'est le rôle du rapporteur. Vous n'êtes pas là pour faire des commentaires sur les amendements à venir, merci. Avis du gouvernement. Excusez-moi, je pense au greffier que je rencontre quand je me rends dans les juridictions, ils sont ravis. Parce que cette mesure. Elle être. Un soulagement de de leur travail au quotidien ce travail répétitif. Symbolise les greffes, ils ont une surcharge de travail que, que personne ne conteste. On permet de transférer ça au commissaire de justice qui l'accepte pour un coût modique. Et là encore je sais pas pourquoi on tergiverse sur quelque chose qui est au fond simple. L'idée parfois je me dis parfois, mais pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué. On a là la possibilité d'alléger le travail de nos greffier ben allons-y enfin pardon pour cet impératif. Bien. Je vais donc mettre aux voix le 47 et le 138 identique avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre.

En cas de contestation d'une saisie de rémunération. Nous souhaitons ainsi aligner le dispositif prévu à l'article 17 sur les autres dispositions du code de procédure civile de l'exécution qui prévoit que le juge de l'exécution et par principe saisie de contestation par assignation et cela quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d'exécution forcée puisque Madame la rapporteure. Vous m'avez fait par. Par avance de votre avis. Négatif. Je tiens à a insisté sur le fait que nous sommes à ce stade. Comme son nom les lundi devant le juge de l'exécution. C'est-à-dire que il y a d'ores et déjà un titre exécutoire alors que. Lorsqu'on parle de de de requêtes. Le le le demandeur, vous le savez dépose. Une demande en face.

potentiel le défendeur. Bénéficie déjà d'un titre. Il serait vraiment malvenue. Par souci de simplification que je peux que je peux comprendre de saisir le juge de l'exécution. Par par requête. Alors que. Le Le créancier a déjà un titre exécutoire, donc ça serait vraiment paradoxal de procéder. Par par requête alors que le créancier et déjà connus et déjà il. Alors. Le titre exécutoire peut émaner d'une collectivité. Qui peut se tromper. Ça n'est pas un juge. Et donc il faut pouvoir. Effectivement aller dans ces cas-là devant le juge et par simple requête c'est quand même plus simple donc défavorable. L'objectif de la réforme. J'ai déjà dit et je le redirai c'est de simplifier et d'unifier le traitement judiciaire des contestations qui sont portées à l'encontre notamment des mesures d'exécution forcée mobilières devant le juge exécution y compris, y compris les modes les modes de saisine qu'il convient d'unifier. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à cet amendement qui permet cette unification. Oui, pardonnez-moi d'insister mais. C'est vrai que, y compris lorsque le titre émane d'une administration dans une procédure. Qui n'a pas bénéficié du contradictoire mais nous avons en face nous avons. Affaire à un titre exécutoire éviter de prendre l'adversaire par surprise précisément l'assignation et le seul moyen. Efficace. De faire de faire régner le principe du contradictoire et de ne pas prendre. Le créancier un traître, si je puis dire.

Que l'on supprime cette possibilité justement dans des situations qui concerneront à la fois des situations d'urgence et des logiques de de modestie des des demandeurs. Ça me paraît un peu curieux Merci je mais aux voit donc le 255, avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Article 17, qui est pour. Qui est contre. Il est adopté à l'article 18 hein. 238 madame Vogel. Merci monsieur le président, si vous le voulez bien, je propose de présenter les les deux d'affilé. Donc ces deux amendements concernent ce qu'on appelle la procédure de légalisation. La procédure de légalisation. C'est la formalité administrative par laquelle les autorités certifie qu'un document qui a été établi à l'étranger est authentique et peut donc être produit devant les autorités françaises. Un acte de mariage, un diplôme et j'en passe. L'amendement 238, il vise à introduire un délai maximal de réponse des autorités et de poser le principe que le silence vaut acceptation de la légalisation. À partir de, donc un délai de 4 mois pour les autorités étrangères puisque en fait il y a des situations dans lesquelles ce sont les autorités des pays tiers qui sont responsables d'accepter ou non la légalisation. C'est le cas par exemple pour la Guinée pour l'Angola et pour les et les ambassades et services consulaires français dans ces 3 pays sont dans l'incapacité de légaliser les actes publics des autorités de ces pays et ils les renvoient donc vers l'ambassade ou le consulat du pays concerné à Paris et donc la procédure dépend entièrement des États tiers. Et il peut arriver que ses services ne répondent pas pour X ou Y raison ou bien répondent très tard et on peut se retrouver dans des situations où toute la procédure en France est bloqué, tout simplement parce que l'acte n'est pas légaliser. On propose donc aujourd'hui pour les pour les autorités françaises ce délai ces deux mois, on propose pour les autorités tiers qu'il soit porté à quatre mais qu'il y en état de sorte que l'on puisse avancer dans la procédure. Le 237. Il vise totalement autre chose. Il vise à. Associer l'assemblée des Françaises et des Français de l'étranger ou. Aux modalités d'application de de formalités administratives. En réalité, ce sont bien nos compatriotes établis à l'étranger qui ont de l'expérience à en la matière. C'est l'enseignante qui ancienne au lycée français dont on arrive rivaux qui a déjà légalisé son acte de mariage malgache en France c'est le papa au Canada qui a légalisé le diplôme de sa fille pour qu'elle puisse étudier en France et donc c'est les conseillers et conseillères qui connaissent des Français de l'étranger qui connaissent au plus près les difficultés de cette procédure et qui peuvent être. Des aides potentielles mais aussi. Des sources de suggestions d'amélioration pour fluidifier les démarches et aussi pour réduire le risque d'erreur parce que l'histoire du cadre légal de la légalisation ne manque pas d'erreur. Je rappelle que l'ordonnance royale de 1681 est issue la procédure avait été abrogée par erreur par une ordonnance de 2006. Et que la nouvelle base légale a été censuré en 2019 par le Conseil constitutionnel parce qu'elle ne prévoyait pas de voie de recours. Pour faire mieux cette fois nous suggérons donc d'associer à cette décision. Les élus qui connaissent le mieux les situations, c'est-à-dire celles et ceux qui sont élus à l'assemblée des Françaises et des Français de l'étranger. Merci. Avis de la commission sur ces deux amendements. Or la légalisation, fait l'objet de multiples accords bilatéraux 1000 multilatéraux qui ne prévoit pas cette possibilité. Il me semble par ailleurs logique que l'administration se prononce explicitement en particulier sur des sujets qui peuvent intéresser l'état des personnes ou à avoir de multiple répercussions contentieuse. Je précise également qu'en matière administrative les situations visées pourront être traitées par une demande d'abrogation de la décision implicite de rejet. Sur un plan pratique, près de 20.000 actes sont légalisés annuellement un tel volume démontre déjà que les services consulaires sont au rendez-vous de leurs obligations. Le temps d'attente peut être certes plus long en fonction des pays, mais cela se règle dans l'immense majorité des cas par l'envoi d'un rappel enfin, il ne me semble pas opportun de revenir sur une disposition votée exactement en ces termes en 2018. Sur le second par contre hein qui. Visent à. À consulter les Français. L'Assemblée des Français de l'étranger. Effectivement les Français établis hors de France étant les premiers concernés par la légalisation des actes étrangers. Il me semble utile de bénéficier de l'expertise de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sur ce point. Donc ce sera un avis favorable défavorable sur le 1er favorable sur le second. Avis du gouvernement, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le président, madame la sénatrice Vogel. Je suis défavorable au premier amendement que vous déposez le 238 pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être. Explicitée par Madame la rapporteure sur le 2ème. Amendement le 238 le 237 pardon. Le Gouvernement émet un avis défavorable. Vous souhaitez en réalité que l'Assemblée des Français de l'étranger soient consultés sur les actes publics concernés par l'obligation de législation et les modalités de la procédure. dépend à la fois des autorités des pays concernés et des autorités récipiendaires répond à la fois des considérations de réciprocité et à des considérations relevant de la coutume internationale la consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger sur ces questions ne paraît pas de nature à apporter des indications complémentaires à cette analyse, basée sur des considérations essentiellement juridique. Merci. Monsieur le comte dans l'explication de vote. Oui, merci Monsieur le. Président, Monsieur le Ministre. Explications de vote sur le 238. Madame la rapporteur je suis désolée de ne pas être d'accord avec vous parce que, justement lorsqu'il a. Une convention internationale justement lorsqu'il y a un accord bilatéral. Le plus souvent c'est pour éviter la légalisation. Donc en réalité nous hein. La légalisation intervient lorsqu'il n'y a pas ces accords là. Or, dans un certain nombre de cas, vous avez des situations où faute de légalisation. D'un acte d'état civil. Les personnes sont en attente parfois plusieurs années d'un document d'identité ce qui est une atteinte profonde à leurs droits et nous pouvons vous en donnez-nous sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger une liste très longue de ces de ces manquements. C'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable de trouver une solution, même si j'ajouterai que. Nous avons dans un certain nombre de cas, la directive donc règle documents publics dans l'Union européenne qui permet d'éviter la légalisation. Et que monsieur le garde des Sceaux. Il est absolument indispensable. Monsieur le garde des Sceaux s'il vous plaît. Il est absolument indispensable que la France revienne dans la commission internationale de l'état civil. Qui permet grâce à un certain nombre de conventions des reconnaissances d'actes d'état civil sans avoir besoin de par la par la les de de de de légalisation. Or la France a quitté la commission internationale de l'état civil qui est pourtant une organisation internationale dont le siège est à Strasbourg c'est c'est particulièrement malheureux et ça bloque un certain nombre d'opérations. pour ce qui est de cet amendement. Je crois qu'il est absolument indispensable de trouver une solution dans les pays pour lesquels ça bouge. Ça ça ça bloque et pour lequel nous ne pouvons pas avoir de légalisation des actes d'état civil et donc souvent. Des droits qui sont bloqués et nous ne pouvons pas nous concentrons-nous nous contenter de. D'attendre des années et des années sans que ça bouge. Voilà donc c'est la raison pour laquelle il est absolument indispensable d'adopter l'amendement 238 et cantons de 137 monsieur le garde des Sceaux. J'ai en tête. Une autre, un autre sujet assez similaire ce sont les les les certificats d'existence pour les personnes qui sont les pensionnés français qui vivent à l'étranger rentre je je fais une à une explication de vote sur le deuxième oui mais vous n'avez pas redemandé la parole donc bon alors ça pas du. Merci et je mets d'abord aux voix puisqu'ils sont pas en discussion commune le 238 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté sur le 237, finissait, Monsieur le comte. Si monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux. Oui, j'ai en tête. Les les certificats d'existence pour les pensionnés français qui vivent à l'étranger. Vous avez raison, ça relève de relations entre les Toutefois, la vie des conseillers des Français de l'étranger et pratiquement utile. Cela n'a pas été fait dans le cas des certificats d'existence et cela révèle dans un certain nombre de pays des choix qui sont inopérants dans la réalité et qui bloquent les personnes dans la capacité d'avoir leur certificat d'existence et nous craignons. Si nous n'avons pas cette consultation pour des raisons d'efficacité et de de confrontation de ce qui est écrit dans les textes avec la réalité. Seuls ceux qui pratique les choses sont capables de le faire que s'il n'y a pas assez de consultation vous avez écrit des choses qui seront dans un certain nombre de pays décalé par rapport à la réalité. C'est la raison pour laquelle une consultation finalement qui ne vaut que par la consultation mais c'est aussi aller chercher des compétences là où elles sont n'est pas inutile et c'est la raison pour laquelle ça vaut la peine de voter cet amendement. Nous allons voir le 237 donc avec un avis favorable. De la commission défavorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est pour.

Que. Compte tenu de la censure partielle des dispositions relatives à la légalisation. La la situation. Qui sortirait du texte issu du Sénat. Si nous ne que le corrigeant pas peut encore poser des risques constitutionnels dans la mesure où justement la censure partielle avait pas de. De mesures. De de de de de de recours contre un refus de de légalisation. C'est la raison pour laquelle nous considérons que fixer un certain nombre de ses modalités, par décret alors que ça devrait être de la compétence du législateur porte encore un risque d'inconstitutionnalité et nous hein vous interrogeant monsieur le garde des Sceaux par cet amendement. Sur ce point et j'en profite, compte tenu d'une modification de l'article 18 dans par nos rapporteurs pour vous demander monsieur le garde des Sceaux. Si vous trouvez opportun. Vous n'avez pas déposer d'amendement que les refus de légalisation relatifs à des documents d'état civil soit porté non pas devant une tribune administratif mais devant la juridiction judiciaire ça nous interroge aussi sur. Un certain nombre de pratiques et de de de tribunal administratif enfin monsieur le garde des Sceaux, j'aimerais avoir une réponse sur la question de la place de la France à la commission internationale de l'état civil, que j'ai évoqué tout à l'heure, merci. Merci avait de la commission. Alors personnellement je ne répondrai que sur l'amendement. Pour dire que je ne partage pas votre analyse qui consiste à dire que les modalités de légalisation d'un acte public étranger ne peuvent être fixé par voie réglementaire puisque. En fait, en 2018, ça s'est bien fait par par voie réglementaire et le Conseil constitutionnel, son problème c'était juste qu'il n'y avait pas de voie de recours. Pas du tout parce que c'était par voie réglementaire. Donc à partir de là. C'est un avis défavorable. Avis du gouvernement. Même position merci je mais aux voix le 48. Monsieur le comte. monsieur le président que je voudrais monsieur le garde des Sceaux apprécié vos réponses sur le fond à une question importante. Je vous rappelle que, si on revient sur ce sujet, c'est parce qu'une censure partielle du Conseil constitutionnel, il me semble que les questions que je pose. Sur les 3 questions posées méritait réponse et je vous remercie de votre exhaustivité.

Oui, merci Monsieur le Président. Alors c'est un amendement d'appel qui. Vise à demander au gouvernement à ce qu'une information claire et accessible présente pour chaque pays et territoires, les obligations en matière de légalisation des actes publics. J'avais jamais regardé pour être honnête. Avant d'étudier ce projet de loi. Le tableau que le ministère produit. Pour la légalisation des actes une ligne pour chaque pays et territoires des colonnes en chiffres Romains et dans chaque cellule une abréviation. Et je vous jure quand vous regardez le tableau. Vous comprenez rien et même quand on a compris à quoi correspondent les chiffres Romains généralement on ne comprend pas quels documents il faut ou non faire légaliser par quelle procédure et. Le problème c'est que comme ce, ce document est très peu compréhensible. On a des sites internet privés qui se sont développées et qui vise à expliquer de façon un peu plus clair. Quel type de document, il faut légaliser dans quel pays avec un outil interactif et des cases à cocher et Ce qui compte. Y a un risque puisque ces sites privés n'ont pas toujours les dernières informations. Et peuvent induire les personnes en erreur donc. Je vais retirer cet amendement mais je voulais juste invité le ministre allemand. Si on pouvait faire quelque chose pour juste quand on cherche l'information. On trouve quelque chose de propret clair dans lequel on s'y retrouve et qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à des sites privés dont l'information est pas toujours à jour. Je vous remercie. L'article 18 qui est pour. Qui est contre. L'article 18 est adopté. Article 19, le 141 monsieur Bena Roche. Oui, monsieur le président. Le présent amendement a pour objet. De s'interroger de s'opposer à la hausse du niveau de qualification pour accéder au concours d'entrée à l'école des avocats. Cette proposition repose sur une volonté d'alignement sur la réforme des diplômes de l'enseignement supérieur LMD mais sans examen de répercussions réelles sur des étudiants, puisque. La sélection drastique opérée pour l'entrée en master deux. Prive de nombreux étudiants en droit d'une poursuite de leurs études vers le master deux et les priverait donc de ce fait également de la possibilité de présenter le concours d'accès à l'école des avocats. De plus, cette réforme imposerait une année d'études soit supplémentaires ce qui pourrait conduire à fermer l'accès à la profession d'avocat aux étudiants les moins aisés. En fait les élèves avocats 108% à tenir un master 1 et effectuent leur master deux après la réussite du concours. CRFPA. Pour laisser plus de souplesse et maintenir une diversité des profils. Il est nécessaire de laisser le seuil du master. Pour la présentation du concours d'entrée à l'école des avocats. Alors en fait le le texte que nous étudions ne défini que le niveau de diplôme pour exercer la profession d'avocat et qui est un master 2. Et effectivement le décret qui prévoit les niveaux de formation ne dissocie pas le niveau de formation pour rentrer au centre de formation et pour exercer la profession d'avocat. Nous avons bien entendu ces remarques. Nous savons que ça touche un nombre non négligeable même s'il est pas énorme mais d'étudiants qui rentrent en centre de formation avec juste un master un et qui passe le master deux avant d'exercer autant il nous sommes nécessaire d'avoir le master de, de telle sorte qu'on aligne à peu près les professions du droit. Sur le Master de par contre effectivement nous demandons mais là c'est vraiment du réglementaire au gouvernement de bien vouloir modifier son décret

j'aurais aimé jusqu'. Le ministre nous dit si si il est prêt à changer le décret quoi puisque c'est l'interrogation que nous nous posons. S'il est prêt à le faire, moi je veux bien retirer la abonnement voilà ben s'il n'est pas prêt à le faire, on va le on va le voter. Donc je mets aux voix le 141. Avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Cet amendement vise à aligner le droit français sur le droit de l'Union européenne en prenant en compte l'expérience professionnelle acquise dans un État membre de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à la profession d'avocat en France les critères d'accès mettent l'accent sur l'obtention un diplôme pour contrebalancer cette préférence notre amendement propose d'inclure l'expérience professionnelle acquise dans un pays membre de de l'UE ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette proposition s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation de la Cour de justice de l'Union européenne qui reconnaissent la validité de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger.

Qui est contre. Il est adopté. Le 49. Madame de La Gontrie. Défendu. Avis de la commission. Même commentaire que précédemment et donc défavorable mais peut-être Monsieur le Ministre va nous répondre sur son sa modification du décret. Monsieur le Ministre. On y travaille. On a entendu. Évidemment ce que vous nous avez dit et on y est pas insensible. Ce qui veut dire que pour le moment c'est un avis défavorable sur l'amendement monsieur le garde des Sceaux. Oui d'accord. Donc le 49 2 avis défavorable qui est pour.

Ce que nous ne souhaitons pas dans cet amendement et ce que l'on souhaite, ce que nous ne souhaitons pas, c'est revenir sur des débats. Entre la profession de juristes d'entreprise et d'avocats et nous ne souhaitons pas plus revenir sur le les débats qui ont concerné profession d'avocat sur le secret de professionnel et donc il n'est pas question. De donner des éléments. À la profession de juriste d'entreprise qui irait au-delà de ce qui a pu être faite pour la profession d'avocat, ce que nous souhaitons, par contre c'est pouvoir préserver la responsabilité des juristes d'entreprise. S'ils étaient mis en cause dans. Le cadre de leur travail de leur mission dite de mise à neuf de la conformité puisque là vous êtes amené à examiner la conformité de la situation de votre entreprise par rapport à votre droit national mais par rapport également à d'autres normes juridiques, en particulier celle d'autres pays dans lesquels l'entreprise exercerait son activité. C'est donc un exercice délicat. Il nous semble que. Le, les derniers mots du premier alinéa c'est-à-dire qui prévoit effectivement une modalité particulière de protection de confidentialité dans la mission de mise en oeuvre de la conformité permettent de bien. Cantonné le. Sujet. Est. De permettre effectivement à cette heure le moment être admis. Si nous avions eu une incompréhension de la portée de ses démons. Nous serons attentifs à écouter le point de vue avec mes collègues de Madame la rapporteur comme du garde des Madame la rapporteur. C'est un sujet important en lien avec l'attractivité de la place de Paris qui avait fait l'objet de recommandations lors des états généraux, ce sera donc un avis favorable. Monsieur le garde des Sceaux. C'est non seulement un sujet important mais c'est également, je suis président, Monsieur le Sénateur, Bonnecarrere. Un sujet difficile. Bon, les entreprises françaises ont sont soumises à des obligations de conformité plus en plus exigeante. Et à défaut d'être protégé par des règles de confidentialité. Les juristes d'entreprise sont. Dans le cadre de leur mission. Mise en difficulté pour élaborer des stratégies internes. Et souvent d'ailleurs ils ont plus de leurs analyses écrites. Et se contentent d'alerter oralement les cadres. Dirigeants s'autocensurent, d'une certaine façon ils sont dans une situation qui est. Très paradoxal ne se fait de voir mettre en oeuvre des obligations de conformité de plus en plus nombreuses alerter les cadres dirigeants des risques juridiques tout en auto-incriminant pas leur entreprise. Tu as un exercice d'équilibriste. Cette situation singulière à l'évidence ne favorise pas la santé juridique et économique de nos entreprises et je pense qu'elle nuit également à l'attractivité de la France, de nombreuses, nombreuses, trop nombreuses directions juridiques choisissent de s'établir dans des pays qui bénéficient de ce les le privilège. Partir du moment, la direction juridique est à l'étranger. Le choix du droit des contrats de l'entreprise sera celui d'un droit étranger. Et donc c'est une question d'attractivité de notre droit évidemment qui est posé. C'est pas une question purement juridique. Derrière le choix du droit applicable. Il y a évidemment des emplois et il y a de l'activité de l'attractivité économique. Et je suis favorable à aménager la confidentialité des consultations juridiques établies par les juristes d'entreprise néanmoins. Néanmoins le bénéfice de cette confidentialité ne peut être accordé qu'à des juristes d'entreprises qui justifie d'un niveau minimal. De diplômes et d'une formation déontologie. Ces éléments sont de nature à s'assurer de la compétence du juriste concernés et de son éthique professionnelle. Bien évidemment, ces mesures ne s'appliquent pas aux matières pénales et fiscales. Je suis favorable à cet amendement. Mais il faut encore. Le retravailler si vous me. Permettez cette. Formulation monsieur le sénateur. Madame de La Gontrie. Pour une explication de vote parce que j'écoute le garde des Sceaux et au fond ce juriste d'entreprise donc être avocat. Comme ça ils bénéficieront du secret. Hé oui c'est quand même des débats qui nous agitent depuis fort longtemps. Donc, personnellement. Nous ne sommes pas favorables à cet amendement. Je comprends bien monsieur le garde des Sceaux que pour le moment, vous êtes favorable à l'amendement. D'accord. Je mais aux voix le 212 avec 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Je mais aux voix l'article 19 qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 20 qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance elle sera reprise à 14h 35 pour la suite de l'examen de ce texte là.